Par courrier en date du mardi 24 octobre 2017, M. Claude Malhuret a informé M. le président du Sénat du changement de dénomination du groupe qu'il préside et qui s'appelle désormais : « Les Indépendants - République et Territoires ». Acte est donné de cette communication. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 et de l'article 56 de la Constitution, la commission des lois a fait connaître qu'elle avait émis, lors de sa réunion du mercredi 25 octobre 2017, un vote favorable- 39 voix pour, 1 voix contre et 1 bulletin blanc -à la nomination de Mme Dominique Lottin aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel. Mme Agnès Canayer, élue juge titulaire à la Cour de justice de la République le 18 octobre dernier, va être appelée à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Je vais donner lecture de la formule du serment. Je vous prie, madame Canayer, de bien vouloir vous lever et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure ». Voici la formule du serment Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui. L'ordre du jour appelle le débat : « Intelligence artificielle, enjeux économiques et cadres légaux », organisé à la demande du groupe Les Indépendants - République et Territoires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la troisième révolution industrielle, celle des technologies NBIC- nano, bio, informatique et sciences cognitives -a commencé en même temps que ce siècle. Elle ne ressemblera pas aux deux précédentes, celle de la machine à vapeur au XIX siècle et celle de l'électricité, du pétrole, des transports et des communications au XX siècle. En effet, son objet est non plus la maîtrise de la matière inanimée, mais la transformation de notre biologie, de notre génome et de notre intelligence, c'est-à-dire tout simplement de l'homme, tout en dotant les machines d'une intelligence et d'une autonomie propres. C'est le défi de l'intelligence artificielle. Ce défi en entraîne beaucoup d'autres. Le premier est économique, et il est alarmant. Pour la première fois depuis deux siècles, la France et l'Europe non seulement ne sont pas à l'origine de cette révolution, mais sont tellement distancées que leur retard peut désormais paraître irrattrapable. Les États-Unis avec les GAFAM- Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft -et la Chine avec les BATX- Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi -sont désormais en situation de duopole au niveau mondial. Pas un seul acteur européen ne s'en approche, même de très loin Au cours des six derniers mois, le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises son intention de redéfinir en profondeur nos politiques numériques. Vous avez vous-même, monsieur le secrétaire d'État, dressé une feuille de route en dix points, qui comporte notamment la couverture numérique complète du territoire et la création d'un fonds de soutien de 10 milliards d'euros dédié à l'innovation de rupture. En juin dernier, au salon Viva Tech, le Président de la République a précisé ses ambitions en matière d'engagement de la France dans ces chantiers « d'innovation de rupture ». L'internet des objets, l'intelligence artificielle, le développement des et sont autant de perspectives prometteuses pour l'industrie française. Ces initiatives sont de puissants gisements d'emplois et de richesses pour notre pays. À l'heure où nous parlons, Angers accueille la 22 édition du, le Salon mondial de l'électronique, de retour en Europe pour la première fois depuis 2005. Je crois que vous y participerez dans deux jours, monsieur le secrétaire d'État. Cette édition française du rendez-vous mondial des leaders de l'électronique pose la question de savoir si notre pays a encore un rôle à jouer dans l'aventure numérique, si nos territoires peuvent faire partie de la dynamique mondiale des nouvelles technologies et si nous pouvons rattraper notre retard. Elle nous invite aussi, en tant que décideurs politiques, à penser cette révolution numérique avant que le vide juridique entourant ces nouvelles technologies ne nous dépasse. Le deuxième défi est social. Contrairement aux prédictions pessimistes qui ont accompagné les deux premières révolutions industrielles, celles-ci, loin d'avoir supprimé des emplois, en ont au contraire créé par millions. De nombreux experts pensent qu'il risque de ne pas en être de même aujourd'hui et que l'automatisation est désormais susceptible de détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée. Ils pensent surtout qu'elle est susceptible de créer un marché du travail à deux vitesses : une minorité d'emplois très qualifiés pour une élite surdiplômée, innovante et maîtrisant les nouveaux codes et une majorité de travailleurs précaires dont les compétences ne rapporteront pas assez pour vivre, sans parler du chômage créé par la substitution pure et simple des logiciels aux emplois les moins qualifiés.

ne seront donc pas les seuls à voir leur travail remplacé partout par la voiture, le train ou le camion autopilotés. Cela nous amène directement au troisième défi, qui est sans doute le plus redoutable, celui de l'éducation. Le plus redoutable notamment pour notre pays, car la naissance de l'intelligence artificielle coïncide avec une chute brutale depuis deux décennies de la France dans tous les classements internationaux, qu'il s'agisse de l'école primaire, de l'enseignement secondaire ou de l'université, qu'il s'agisse de l'enseignement des mathématiques, qu'il s'agisse de l'enseignement des mathématiques, de la langue maternelle ou des langues étrangères ou encore qu'il s'agisse de la montée des inégalités dans l'accès à la connaissance. C'est au moment où l'école va devoir affronter le rendez-vous d'une remise en cause et d'une adaptation drastique au monde nouveau des logiciels que notre pays s'y présente en situation d'extrême faiblesse. La question est simple : l'éducation nationale française est-elle aujourd'hui susceptible d'aborder dans de bonnes conditions la révolution du développement des compétences qui seront de plus en plus transmises par les nouvelles technologies ? À première vue, la réponse paraît négative. Il semble bien que le nouveau ministre de l'éducation nationale soit fort conscient de ce problème, mais quel défi va-t-il lui falloir relever !

Cette éducation nationale qui n'est pas aujourd'hui en grande forme va devoir, en plus de son rôle actuel, former des enfants et des adolescents à vivre dans un monde où intelligences biologiques et artificielles devront cohabiter, et cela avec un corps enseignant qui, dans son immense majorité, et ce n'est un secret pour personne, ne maîtrise pas encore lui-même les nouvelles technologies. Le quatrième défi est juridique et pose mille questions différentes, inédites et, la plupart du temps, contradictoires.

sur l'assignation de responsabilité en cas d'accident d'un véhicule autonome ? Il y a des milliers de questions comme celles-là ! La loi du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils nous a permis de nous engager dans ce débat de la responsabilité de l'intelligence artificielle et des robots.

d'accompagner le développement de ces technologies. Enfin, le dernier défi que j'évoquerai, mais il y en a bien d'autres, est peut-être l'un des plus difficiles à relever : c'est celui de l'éthique et de la morale. Il se pose dès aujourd'hui. Toutes les applications en faveur de la santé ou de la préservation de la vie interrogent très fortement sur le respect de la vie privée. Comment s'assurer que ces données de santé ne seront pas vendues à une compagnie privée ou à un futur employeur ? Comment conjuguer cette collecte massive de données de santé de chaque Français et le respect du « droit à l'oubli » comment s'assurer qu'intelligence artificielle et robotique riment avec traitement des données éthique ? Ce défi se pose dès aujourd'hui, mais il sera encore plus sérieux demain. Franchirons-nous l'étape du transhumanisme, cette idée que l'homme peut être « augmenté » ou « amélioré » par la machine ? Et si nous la franchissons, ce qui est désormais probable et en cours de réalisation, notamment en Chine, un pays évidemment moins soucieux que le nôtre du respect des droits, comment accepter que cette « augmentation » ou cette « amélioration » de l'humain soit réservée à ceux qui pourront en payer les coûts extravagants ? Cet enjeu de l'hybridation de l'homme et du robot ne peut s'envisager sans règles. De même que la recherche sur les cellules souches ou les embryons fait l'objet d'une réglementation forte, le couplage de l'intelligence artificielle et de l'homme doit être encadré par un texte précis. La transformation du corps humain sous l'effet de l'intelligence artificielle est un sujet radical, sur lequel un débat public doit être mené en y associant l'ensemble des parties prenantes. Je parlais des défis éthiques d'aujourd'hui et de demain, mais ils ne sont rien par rapport aux défis d'après-demain, lorsqu'apparaîtra l'intelligence artificielle dite « forte » dotée de conscience, mais inscrite sur un support de silicone et non plus sur le support organique de notre ADN et de notre cerveau. Ce jour-là- il n'est heureusement pas encore à l'horizon, mais il arrivera -, nous devrons décider si nous permettons, pour reprendre la très belle phrase de Michel Foucault à la fin des, que la figure de l'homme s'efface peu à peu, « comme à la limite de la mer un visage de sable Et même si cette décision est une affaire de plusieurs décennies, peut-être vaut-il mieux commencer à y réfléchir dès maintenant. Il reste un dernier problème à aborder, celui de la dimension européenne du sujet. L'Europe est confrontée à un dilemme fondamental qui n'est pas résolu et qui la place dans une situation intenable face à ses concurrents américains et chinois. Elle a donné jusque-là la priorité à la protection des citoyens quant à l'utilisation qui peut être faite des données les concernant. Cette position nous paraît une évidence, mais il faut bien comprendre qu'une de ses conséquences est le monopole américano-chinois sur l'intelligence artificielle. Peut-on trouver aujourd'hui, et dans le cadre d'une discussion toujours longue et difficile, car nous sommes la juste mesure entre la protection des droits et l'utilisation des données permettant de faire naître chez nous l'équivalent des GAFAM et des BATX ? C'est l'un des enjeux fondamentaux de la place de l'Europe dans le monde de demain et, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. En janvier 2017, le Parlement européen a adopté un projet de résolution de la Commission européenne contenant des recommandations concernant les règles de droit civil sur la robotique. Le législateur européen a notamment mis en place un régime de responsabilité limitée pour les différents acteurs de la filière et un fonds de compensation. Ce sont des engagements forts, que la France doit accompagner. Mes chers collègues, si nous avons choisi d'interpeller aujourd'hui le Gouvernement sur cette question de l'intelligence artificielle, c'est parce que nous estimons qu'elle suscite de formidables occasions, mais pose aussi de profondes questions économiques, sociales, juridiques et éthiques. Il est du devoir du politique d'anticiper ce genre de rupture et de ne pas seulement agir en réaction au quotidien. C'est en réaction au quotidien. C'est la dernière raison pour laquelle, monsieur le secrétaire d'État, le groupe Les Indépendants, soucieux de relever ce pari numérique, souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle et pour mettre en place un cadre juridique et légal national, et bien sûr européen, permettant à notre continent, tout en se protégeant d'éventuelles dérives, de garder son rang dans un monde où le changement ne cesse de s'accélérer. La parole

Un troisième ingrédient de l'accélération est, quant à lui, purement humain. Il s'agit du niveau de recherche en algorithmes et en intelligence artificielle. La source de l'efficacité d'un dispositif d'intelligence artificielle, c'est la capacité de calcul, ce sont les données sensibles, mais c'est aussi l'intelligence des algorithmes.

ailleurs. Je le répète, nous ne sommes pas là pour subir, nous n'avons rien à subir, nous avons tout à décider. Encore faut-il savoir quel chemin nous voulons tracer. Encore faut-il savoir où nous voulons aller. C'est tout l'enjeu de la mission que nous avons confiée à Cédric Villani.

l'enjeu de ce rapport sera non pas d'apporter une réponse en la matière, mais de souligner les questions éthiques que nous devrons offrir aux Français et auxquelles nous nous donnons pour mission de répondre dans les prochains mois.

beaucoup de bon sens. Nous allons maintenant procéder au débat sous forme de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Les auteurs des questions disposent chacun de deux minutes, y compris pour la réplique.

Je prendrai le simple exemple des modes de déplacement des personnes et des marchandises avec les véhicules autonomes, dont on prévoit l'arrivée des premiers exemplaires sur le marché début de 2020, avec une généralisation à partir de 2030. Ces derniers vont remplacer progressivement plusieurs millions de travailleurs : les chauffeurs de poids lourds en premier, puis les chauffeurs de taxis et autres VTC, enfin les chauffeurs de bus et autres transports en commun. Il d'une occasion extraordinaire en termes de sécurité, de confort, de productivité, de diminution des impacts environnementaux. Toutefois, cela crée de profondes inquiétudes. Tout d'abord, dans un marché du travail qui va perdre plusieurs millions d'emplois, lesquels seront remplacés par seulement quelques centaines de milliers d'emplois hautement qualifiés dans les hautes technologies, quels mécanismes devons-nous mettre en place pour partager les richesses créées par cette intelligence artificielle artificielle et financer les nécessaires emplois dans les services publics, notamment ceux qui sont liés à l'aide à la personne, dont on sait que l'on va avoir un besoin croissant avec le vieillissement de la population française et européenne ? Dernière interrogation, que vous avez vous aussi soulignée, sommes-nous en mesure d'impulser les dynamiques nécessaires au niveau national et international afin de traiter de l'ensemble des questions éthiques qui vont se poser de manière aigüe au fur et à mesure des développements de cette intelligence dite « artificielle

coordination entre le calendrier du véhicule autonome et le cadre législatif et réglementaire qui en définira les modes d'usage.

ouverts à tous et permettant à toutes les personnes, en fonction de leur situation géographique et de leur capacité physique, de se déplacer d'un point à un autre pour assurer tous les éléments de la vie. Il y a différentes façons d'atteindre

du minitel et d'internet, je souhaiterais que le pouvoir politique soit modeste et laisse une large place à la fois aux techniciens, aux scientifiques, aux investisseurs, aux consommateurs et aux citoyens. Il ne faut pas

de poser le cadre d'une discussion globale, c'est-à-dire véritablement politique. Si nous voulons construire de bonnes politiques publiques dans le domaine de l'innovation et, en particulier, dans celui de l'intelligence artificielle, il faut se poser certaines questions.

peut-on envisager la régulation de ces développements pour qu'ils ne deviennent pas incontrôlés ? Il se trouve qu'un élément de réponse a été apporté par le Président de la République lors de son grand discours sur l'Europe, le 26 septembre dernier, à la Sorbonne, à savoir la création d'une agence de l'innovation de rupture. Cette agence qui,

Je vous remercie

Dans un tel cas, nous avons plusieurs outils juridiques à notre disposition. Il y a, tout d'abord, la standardisation des protocoles, qui vise au moins à s'assurer que les différents véhicules autonomes parlent le même langage et que, dans notre ville connectée, ils puissent échanger les uns avec les autres. délégation de service public pour l'infrastructure et la partie profonde du réseau. Qu'est-ce qui fera fonctionner les voitures autonomes de demain ? À l'heure de l'intelligence artificielle et de l'autonomie énergétique, ces réseaux ne sont pas forcément physiques. Cela pose une question très actuelle pour le Gouvernement : est-il du rôle des collectivités locales

L'accroissement rapide et imprévisible des tâches potentiellement automatisables nous amène à nous interroger sur les activités humaines futures. On passe d'un système où les emplois très manuels et ceux qui sont fondés sur les talents semblaient préservés de l'automatisation à un scénario de transformation qui touche potentiellement beaucoup plus de monde. Ainsi, selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, ou COE, la destruction d'emplois pourrait être moins étendue que nous le pensons et se chiffrer à moins de 10 % des emplois. l'automatisation entraînerait une transformation importante d'un emploi sur deux. En effet, d'après un rapport du Conseil national du numérique de mars 2017 visant à anticiper les impacts économiques et sociaux de l'intelligence artificielle, les conséquences seraient « moins destructrices que transformatrices du travail Le but à atteindre est de créer de la valeur dans le travail pour toutes et tous, de donner plus de pouvoir et d'intelligence et non pas de mécaniser les humains. Les politiques publiques, nationales et régionales, doivent être mobilisées pour construire une vision positive de l'intelligence artificielle, ce qui nécessite de placer la formation au coeur du travail. En cela, l'intelligence artificielle rejoint notre projet « sécurité emploi-formation », qui vise à permettre à chaque travailleuse et à chaque travailleur d'alterner emplois stables et correctement rémunérés et formations permettant d'accéder à de nouveaux emplois. L'intelligence artificielle peut soit provoquer une hémorragie des emplois dans certains secteurs professionnels, soit, au travers d'une redistribution des gains de productivité, financer des formations évolutives et une montée en gamme des qualifications. Tout dépend de la volonté politique. Monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous d'accord pour que l'on utilise l'intelligence artificielle afin de libérer le salarié du travail fastidieux et répétitif, en réduisant la charge et le temps de travail ? Monsieur le sénateur, vous abordez plusieurs questions : la transformation du travail, les économies liées à l'intelligence artificielle et la capacité que nous aurons à la maîtriser. Vous avez cité le rapport du COE et évoqué celui du Conseil national du numérique, qui a été rendu à l'époque où j'en étais le président.

en introduction. On soulignera, avant tout, que, au niveau français comme à l'échelle européenne, nous n'avons, hélas, ni l'ambition ni la stratégie pour une véritable politique industrielle des nouvelles technologies. Alors que nous devrions concentrer tous nos efforts sur le développement et l'ancrage européen de notre écosystème technologique, nous assistons à une hémorragie des talents et de nos start-up, rachetées par des groupes américains ou asiatiques. Soyons lucides : il s'agit bien d'une guerre d'intelligence économique. Le traitement en masse des données et les algorithmes de l'intelligence artificielle sont en effet devenus des enjeux stratégiques pour notre économie et notre défense. Toutes les nations qui ont développé des écosystèmes technologiques puissants l'ont fait grâce à des politiques volontaristes. Les Américains ont orienté, dès 1953, leur commande publique vers les PME grâce au. Cela a permis aux Cela a permis aux PME américaines innovantes d'obtenir d'emblée des contrats fédéraux ou locaux. Ces mécanismes d'achats et d'aides publiques intelligentes sont à l'origine des plus grandes réussites américaines, comme celle d'Elon Musk avec Tesla. Ces géants technologiques se sont aussi développés grâce à des exemptions fiscales et à des mesures d'aides gouvernementales. Il n'y a d'ailleurs pas une seule des technologies clefs de l'iPhone qui n'ait été, à un moment ou un autre, subventionnée par l'État américain. Plutôt que d'établir de grands plans industriels souvent inefficaces et qui se résument trop fréquemment à du saupoudrage vers les grands groupes, l'État doit absolument innover et contribuer à faire évoluer la réglementation européenne de la concurrence. contre-productive : elle ne permet pas à nos PME de devenir des entreprises de taille intermédiaire, puis des acteurs internationaux. Tel est bien l'enjeu à ce moment clef où nous mesurons le potentiel, mais aussi les risques, que recèle l'intelligence artificielle. Aussi ma question est-elle simple ; elle rejoint

l'échelon national, d'identifier ces technologies de rupture ; en effet, on peut toujours appeler à la création d'un fonds pour l'investissement dans les technologies de rupture, mais encore faut-il les identifier. Les pays que vous avez cités, ceux qui ont réussi à avancer sur ces sujets, pilotent, au niveau régional ou national,

Comment, et à quel niveau financier, le Gouvernement prévoit-il d'accompagner la recherche et le développement de l'intelligence artificielle dès le projet de loi de finances pour 2018 et au cours des années suivantes ? Je note par ailleurs que, dans ce rapport, l'agriculture n'est pas évoquée. évoquée. L'intelligence artificielle se prêterait pourtant bien à l'assistance de nos agriculteurs en matière de pilotage et de stratégie d'exploitation. La constitution et l'exploitation d'un agricole auraient des vertus multiples, y compris en matière de simplification administrative pour les agriculteurs. Qu'est-ce que le Gouvernement se propose de faire ou d'impulser en la matière ? Pour finir, comment le Gouvernement entend-il donner une chance aux territoires hors métropoles pour contribuer au développement de l'industrie de l'intelligence artificielle Comment associer les villes moyennes aux écosystèmes créatifs en question ?

d'une compétition internationale de start-up dirigées par des femmes. La lauréate avait développé une technologie d'intelligence artificielle dans la personnalisation et l'identification de soins contre le cancer. Sa start-up

la vie digitale, l'industrie 4.0 ou l'écosystème numérique français. Vous y serez demain et après-demain, monsieur le secrétaire d'État, et le Premier ministre y viendra vendredi. aura fallu, vous l'avez dit, un combat de plusieurs années, sinon de plusieurs décennies, ainsi qu'une volonté politique forte, pour faire venir ces décideurs en Anjou, sur notre territoire, et mettre ainsi en valeur nos savoir-faire. C'est aussi l'accompagnement et le développement des réseaux dans le monde entier. Nous devons continuer à développer ces nouvelles technologies en nous appuyant sur notre filière industrielle d'excellence.

Notre pays doit rapidement s'engager dans une stratégie de souveraineté numérique. Cette dynamique peut d'ailleurs trouver un écho à l'échelon européen, comme l'a rappelé Claude Malhuret. Ma question est simple quelle est la volonté du Gouvernement et quels sont les moyens accordés par l'État à la défense de notre souveraineté numérique et au développement d'une filière industrielle française de l'intelligence artificielle ?

la valorisation de titres déjà détenus dans d'autres entreprises. Cette somme, constituée en fonds, nous permettra de mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros par an sur les fameuses technologies de rupture,

de notre pays. Les technologies fondées sur l'intelligence artificielle, dont l'apparition remonte déjà au milieu du XX siècle, monsieur le secrétaire d'État, ont des effets substantiels tant sur les individus que sur l'économie et la société. Porteuses d'innovations fascinantes, elles posent des problèmes résultant de leur intégration au sein des « systèmes institutionnels » et suscitent aussi de vives inquiétudes en matière d'éthique, mais aussi et surtout d'emploi. Tous les pays ne jouent pas à armes égales. En Suède, près de 6 % des salariés travaillent dans le secteur de la communication électronique, contre seulement 1,2 % en Grèce. La France, quant à elle, est dans la moyenne européenne, avec 3,6 %. Lancée à la fin du mois de janvier, l'opération « France IA » a mis en place dix-sept groupes de travail mobilisant quelque cinq cents experts, chercheurs et représentants du monde de l'entreprise chargés de définir une stratégie de mise en valeur et de développement de cette filière.

S'il est vrai que les recherches actuelles en sciences économiques ne permettent pas encore d'apprécier précisément les effets de l'IA, elles pointent néanmoins les risques de destruction d'emplois ou de dénaturation des emplois Permettez-moi dans ce cadre, monsieur le secrétaire d'État, de faire un parallèle avec le plan pour la formation professionnelle présenté récemment par le Président de la République. Ma question est simple : les politiques publiques envisagées sont-elles suffisamment attractives pour permettre à ceux qui en auront besoin de se former ou de se reconvertir grâce à la filière de formation nationale sur l'intelligence artificielle ? La parole est

avons décidé d'avoir une vision très pragmatique, qui traite à tous les étages des différents niveaux de compétences. Ce sont d'abord les compétences numériques universelles, ou « littératie numérique », qui doivent être accessibles à tous

semblent une évidence pour nous tous, mais qui, aujourd'hui, ne sont pas maîtrisées par près de 13 millions de Français, soit quasiment 20 % de la population.

au sein d'une : j'ai dépanné près de 9 000 Français au téléphone et je me fais une fierté d'avoir été de ceux qui accompagnent nos concitoyens à maîtriser les technologies. Je veux qu'il y en ait encore plus en France.

Notre pays dispose d'importants atouts à faire valoir dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle. Certes, les États-Unis ou la Chine sont réputés être les pays les plus avancés, mais nous nous en sortons plutôt bien. Les applications de l'intelligence artificielle peuvent concerner l'éducation, l'environnement, les transports, l'agriculture, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les applications pour l'aéronautique, la sécurité et surtout la défense : oui, de nouvelles perspectives s'ouvrent en matière de défense avec l'intelligence artificielle. Le rapport Gillot-de Ganay préconise d'encourager la constitution de champions européens en intelligence artificielle et en robotique, tout en poursuivant le soutien aux PME spécialisées, en particulier les start-ups. J'aimerais prolonger ce point par ma question. Nous assistons à domination de quelques entreprises, le plus souvent américaines, parfois chinoises, concernant l'intelligence artificielle. Je pense aux GAFA, qui représentent la pointe de la recherche, mais la Chine, avec les BATX, veille au grain. le secrétaire d'État, quelle place existe pour l'Europe et pour la France ? Quelles initiatives ou mesures le Gouvernement entend-il prendre pour contribuer à l'émergence de champions européens en intelligence artificielle ? J'en arrive à ma question sur la défense. Comment le Gouvernement conçoit-il le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans le secteur de la défense ? Quels projets envisage-t-il par exemple de soutenir pour favoriser des applications d'intelligence artificielle dans ce secteur ? La parole

aujourd'hui, nous avons un déficit de fournisseurs européens d'éléments matériels centraux dans nos réseaux, ce qui entraîne notre dépendance à l'égard de fournisseurs venus d'autres continents. Dans le domaine de la défense, c'est encore plus essentiel, puisque nous sommes l'une des grandes nations qui participent

Nos collègues Dominique Gillot et Claude de Ganay ont rendu au mois de mars dernier, sur l'initiative de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un copieux rapport sur l'intelligence artificielle. Sans que le bilan qu'ils dressent et les perspectives qu'ils proposent aient été réellement discutés, le Gouvernement a demandé à M. Cédric Villani un nouveau rapport sur le sujet, moins de six mois après le dépôt du précédent. M. Cédric Villani est par ailleurs président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques : vous nous permettrez par conséquent de nous interroger sur le bien-fondé de ce cumul, qui nous semble déontologiquement discutable. À l'occasion de ses nombreux entretiens avec la presse, M. Cédric Villani défend une approche globale de l'intelligence artificielle et, sur ce sujet, nous ne pouvons que partager son point de vue. Il nous semble, en effet, que ce dossier ne peut être dissocié des difficultés rencontrées par la culture mathématique, singulièrement par son apprentissage scolaire. Pour n'en donner que quelques exemples, je rappelle qu'un quart des collégiens ont des difficultés en mathématiques. Pis, sur les 1 440 postes ouverts au CAPES de mathématiques, 375 sont restés vacants. De nouveau, cette année, depuis la rentrée, nous entendons dans nos départements la récurrente plainte des familles exaspérées par le non-remplacement des professeurs, qui touche principalement les disciplines scientifiques. Ne pensez-vous pas qu'une stratégie efficace en matière d'intelligence artificielle devrait en tout premier lieu renforcer la culture scientifique dans l'enseignement ? Par ailleurs, le rapport de Dominique Gillot et Claude de Ganay faisait justement apparaître la nature essentiellement masculine de la recherche en intelligence artificielle. Environ 90 % des programmeurs et des développeurs sont des hommes. Pourquoi les femmes sont-elles exclues à ce point de ces disciplines ? Par quel processus mystérieux l'intelligence féminine ne pourrait-elle pas se développer dans le domaine de l'intelligence artificielle ? La parole

La question est sans doute l'une des plus importantes du moment. Deux visions s'affrontent aujourd'hui pour y répondre : une vision malthusienne et une vision schumpéterienne. Selon la première, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il n'y aurait pas de destruction créatrice, ce qui semble attesté par certaines études. Par exemple, Frey et Osborne, deux chercheurs d'Oxford, ont estimé en 2013 que la moitié des emplois aux États-Unis seraient remplacés à terme par une machine, au sens large. C'est sur cette vision que se déploient toutes les théories du revenu universel garanti. Cette vision, ce n'est pas la mienne. Certes, la révolution numérique sera aussi fatale aux cols blancs que l'automatisation industrielle l'a été aux cols bleus, mais les cols d'or arrivent, la, comme l'a appelée le professeur de Columbia Richard Florida. C'est aussi l'analyse du spécialiste de l'intelligence artificielle Laurent Alexandre, qui explique que les métiers de demain devront être complémentaires de l'intelligence artificielle. De nouveaux métiers se profilent donc et constituent un fantastique gisement pour l'avenir. Le défi pour la puissance publique est de les identifier pour informer et former. Monsieur le secrétaire d'État, comment notre pays s'y prépare-t-il ? encore une question très large, qui pose peut-être même la question de la question

chacun, avec ses propres compétences, parvient à émerger. À cela s'oppose un autre modèle, dans lequel les champions gagnent tout, les entreprises championnes font émerger en elles-mêmes des

ne crée pas de nouveaux mégamonopoles qui engendreront des monstres économiques, mais aussi des monstres démocratiques ? Quand certaines entreprises dépasseront le million de salariés, ce qui sera possible dans un monde où les structures et les mégaplateformes s'intégreront de façon verticale ou horizontale dans toutes les strates de notre vie économique, ceux qui seront à leur tête poseront des questions sur notre propre pouvoir et sur notre légitimité à décider du sort de leurs citoyens-salariés, qui seront peut-être plus salariés que citoyens, eux qui iront vivre sur des îles flottantes dans les eaux territoriales internationales. On pourra alors se poser des questions.

très rapidement à propos de cette coproduction : que vont devenir les données d'apprentissage fournies par les élèves et les enseignants ? de la notion de propriété intellectuelle, des plateformes coopératives, collaboratives ? Comment

de vérité exacte, juste et nécessaire. Cette capacité à débattre, cette capacité créative à orienter le monde, cette capacité à décider ce qui est souhaitable pour les hommes et peut être aussi pour les machines

Pour le moment, nous assistons au succès des algorithmes de Google et de Facebook, efficaces pour trouver des réponses à nos questions et pour hiérarchiser un certain nombre d'informations. Les chercheurs réalisent des programmes informatiques qui surpassent l'homme dans certaines de ses capacités cognitives. Je pense notamment au jeu d'échecs, au jeu de go ou même au ping-pong ou au poker. Un bon progrès sera celui qui saura bien accompagner l'essor de ces technologies. Il a déjà été rappelé que notre collègue député Claude de Ganay et notre ancienne collègue Dominique Gillot ont rendu,

et Dominique Gillot proposent, par exemple, d'élaborer une charte de l'intelligence artificielle et de la robotique et de confier à un institut national de l'éthique de l'intelligence artificielle et de la robotique un rôle d'animation du débat public sur les principes éthiques qui doivent encadrer ces technologies. Monsieur le secrétaire d'État, au-delà de la mission confiée à notre collègue député Cédric Villani, dont l'intelligence est incontestable,

Quelle qualité d'usage l'intelligence artificielle peut-elle apporter ? On a évoqué les voitures individuelles, mais je suis plus particulièrement attachée, pour ma part, aux transports publics. Les navettes autonomes peuvent transformer radicalement nos politiques de mobilité. Elles ouvrent des perspectives inédites pour garantir une meilleure continuité du service public des transports et permettre ainsi un maillage plus fin du territoire dans l'espace. Notre assemblée ne peut bien évidemment qu'être sensible au potentiel de telles navettes pour desservir les centres-villes historiques et la ruralité. Des navettes de rabattement en zone rurale pour connecter un mode lourd sont d'une grande utilité. Actuellement, on sait très bien que les transports à la demande fonctionnent avec grande difficulté, la navette autonome peut aussi améliorer la continuité du service public dans le temps, avec des transports publics qui fonctionnent à des horaires atypiques, par exemple pour du personnel d'entretien

L'exemple lyonnais de la navette autonome Navly, qui, avec le Sytral et Keolis, fonctionne sur le quai dans le nouveau quartier de la Confluence, est tout à fait intéressant à suivre, mais la réglementation actuelle ne permet pas aux collectivités de mettre en oeuvre librement ces expérimentations. Monsieur le secrétaire d'État, j'imagine que vous réfléchissez déjà à l'adaptation de ce cadre juridique avec votre collègue Élisabeth Borne. Plus globalement, comment les Assises de la mobilité et le projet de loi d'orientation qui en découlera prendront-ils en compte cette évolution technologique majeure ? On nous permettra d'innover dans nos territoires, d'exercer le droit à l'expérimentation, ainsi que le droit à l'erreur.

que les modalités de transport que nous utilisons pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes malades, les collégiens ou les lycéens sont des systèmes imparfaits,

Gleut. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'intelligence artificielle va totalement révolutionner nos vies et encore davantage celle de nos enfants. L'intelligence artificielle va, par ailleurs, totalement révolutionner le marché de l'emploi. Il se trouve que les leaders mondiaux sont les GAFA américains- Google, Amazon, Facebook, Apple -et les BATX chinois-

une véritable industrie de l'intelligence artificielle française, avec des acteurs privés français, dans une combinaison avec le travail de l'action publique ? La parole

l'État, la DINSIC, qui est acteur de la transformation numérique de l'État, avec une équipe technologique que j'ai renforcée, qui va recruter, dans les prochains mois et les prochaines années, des profils de très haut niveau liés aux technologies et à l'innovation appliquées aux domaines d'intervention de l'État et qui travaillera en collaboration avec

J'ai bien compris la volonté des auteurs de ce rapport de démystifier l'intelligence artificielle et de contrer tout fantasme et toute dérive qui consisterait à admettre que l'humain, au XXI siècle, serait, à court ou moyen terme d'ailleurs, supplanté par une intelligence supérieure, un peu à l'image de ce que fut, pour l'homme de Neandertal, l'apparition d'voilà 30 000 ans. Néanmoins, ce rapport évoque des risques, dont la maîtrise ne semble pas complètement assurée. On évoque ainsi, sur le plan technologique, des questions liées à la sûreté, à la sécurité et à la robustesse des systèmes, au phénomène de boîtes noires des algorithmes, de. La régulation englobe la prévention et le contrôle, apparaît d'autant plus nécessaire que des pays comme la Chine, qui investissent massivement dans le secteur, ne semblent pas très proactifs sur la réponse à apporter aux questions d'éthique.

Ma question concerne plus précisément la justice. S'il faut sans doute se garder d'une vision prophétique telle que celle que l'on peut trouver dans l'univers de Philip K. Dick avec, les ont commencé à développer ce que l'on appelle communément un champ de « justice prédictive Dans le débat public, les premiers échos ont résonné autour d'une étude universitaire britannique menée sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Un outil créé pour l'occasion a défini des modèles de jugement et a pris des décisions similaires à celles de la CEDH dans 79 % des cas qui lui ont été soumis. Certains y ont vu la possibilité que des robots remplacent un jour les juges ou les avocats. En réalité, il pourrait davantage s'agir d'un outil permettant de rationaliser certaines étapes de la saisine, un outil utile aux justiciables, aux avocats comme aux juges, et finalement pas si éloigné de nos anciennes bases de données. Pour certains champs très engorgés de la justice, cette justice prédictive permettrait sans doute de favoriser des accords à l'amiable plutôt que des procédures longues et coûteuses dont l'intelligence artificielle prédirait qu'elles trouveraient une issue facile à deviner. Partant de la même vision pragmatique, le législateur a voulu appliquer le principe d'ouverture des données publiques aux décisions de justice administrative et judiciaire dans la loi pour une République numérique. Puis, au printemps dernier, en partenariat avec le ministère de la justice, les cours d'appel de Rennes, en Ille-et-Vilaine, et de Douai, dans le Nord, avaient décidé d'expérimenter une solution de prévisibilité de la justice. Cependant, la semaine dernière, des articles de presse se sont fait écho d'une réception très différenciée entre les cours d'appel de Rennes et de Douai sur ces expérimentations. Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous éclairer la représentation nationale sur la manière dont ces expérimentations progressent et nous rassurer sur la volonté continue du Gouvernement de poursuivre l'ouverture des données publiques

Aujourd'hui, l'enjeu est plutôt d'assister le citoyen, les professionnels de justice, les greffiers et les juges dans le transfert, l'analyse et le traitement de la masse d'informations, plutôt que

: il y a surtout une confiance dans l'outil. les nouvelles formes de technologies, permises par le développement de l'intelligence artificielle, agrémenteront demain le quotidien de chacun, en particulier celui de nos enfants. En effet, les jeunes générations vont grandir avec ces avancées technologiques et de nouveaux comportements et besoins vont apparaître. Des informaticiens, ingénieurs, mathématiciens, voire philosophes vont être nécessaires pour répondre à cette demande. La place de l'intelligence artificielle dans le système éducatif doit être anticipée, soit comme outil complémentaire pour les enseignants, soit comme matière d'enseignement ou de recherche. L'intelligence artificielle permettra donc un saut qualitatif pour aider les personnes en situation de handicap, en proposant des exercices de curiosité et de stratégie, mais aussi pour les élèves, en systématisant les chaînes d'apprentissage pour les exercices de mémoire. Un professeur de mathématiques de ma belle ville de Besançon a mis en place un individuel d'apprentissage du calcul mental, le projet Mathador. L'intelligence artificielle est donc un outil formidable pour accompagner la dimension plus automatique ou systémique que celle, consciente, de l'éducation. Il ne s'agit pas de céder aux sirènes d'un défi quantitatif, mais bien de s'attaquer au qualitatif. La pensée d'Edgar Morin résume cette problématique, car, pour lui, l'enjeu de l'éducation, eu égard à l'intelligence artificielle, n'est pas d'avoir un homme augmenté, mais un homme amélioré. Il y a donc un volet clé, c'est la question des algorithmes, de leur puissance et de leur périmètre d'action. On pourrait se demander quel algorithme en matière de formation ou quel algorithme éducatif se chargera d'éduquer les logiciels éducatifs

Parmi ces dernières, assez proches des apprentissages statistiques, l'apprentissage profond ou, évoqué tout à l'heure, est devenu dominant au cours des dernières décennies, en particulier au cours des quatre dernières années.

la question concernant davantage les données que les algorithmes eux-mêmes. Ces algorithmes reproduisent en effet les biais des données qu'ils traitent, en particulier toutes les discriminations qui existent dans nos sociétés tant qu'elles ne sont pas corrigées.

Dany Wattebled, je vous présenterai une première approche de ce dispositif ancien, aujourd'hui remis au goût du jour. Lors de son intervention télévisée du 15 octobre 2017, le Président de la République a souhaité remettre sur la table des négociations la question de l'intéressement et de la participation des employés aux entreprises françaises. À ce titre, le Président a évoqué une « belle invention gaulliste Ce thème, porté par des gouvernements successifs, est entré partiellement dans notre droit, y compris dans le code du travail. Toutefois, si la participation financière est bien une réalité, à travers les multiples dispositifs d'épargne salariale, il en va différemment de l'autre participation, celle, plus diffuse, plus sociale que Charles de Gaulle évoquait dans son discours devant les mineurs de Saint-Étienne en 1948 : « Dans un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail. » L'ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises n'est qu'un succédané de la pensée gaulliste. C'est une simple étape vers un ordre social nouveau, marqué, lui, par la triple répartition aux bénéfices, au capital et aux responsabilités. En 2015, 8 millions de salariés ont eu accès à au moins un dispositif de participation, d'intéressement ou d'épargne salariale. En effet, la participation est obligatoire pour les entreprises réalisant un bénéfice supérieur à 5 % de capitaux propres. Pour assurer son développement, les gouvernements précédents ont mis en place une exonération de certaines cotisations en cas de blocage des sommes. En contrepartie, à partir de 2008, certaines ont été soumises au forfait social. La loi d'août 2005 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a permis des avancées notables une simplification, avec un renouvellement des modalités de reconduction tacite des accords d'intéressement ; un élargissement, avec le recours à la négociation de branche et la mise en place d'accords d'épargne salariale « clés en main une réforme du financement des PME, avec une modulation à la baisse du forfait social. Affirmer toutefois qu'environ la moitié des salariés bénéficient d'un type de participation financière, c'est reconnaître que la moitié reste à l'écart. Le bilan est donc en demi-teinte. Les déblocages exceptionnels pratiqués dans le passé, dont le dernier sous la présidence de François Hollande, n'ont pas atteint les objectifs de relance et sont perçus comme une menace pour la situation financière des entreprises. Il ne faut pas pour autant baisser les bras. Les maux sont connus et analysés de longue date : la faible connaissance par les salariés des dispositifs, la forte suspicion de fraude ou de détournement. Dès lors, quelles perspectives pour cette belle idée gaulliste ? Est-ce l'extension de la participation obligatoire à toutes les entreprises sans seuil minimal ? Dans son intervention, le chef de l'État semble vouloir construire un nouveau compromis social et politique. Mais que deviendra cette idée dans le futur projet de loi « Entreprises » porté par le ministre de l'économie en 2018 ? La participation et doit être la composante principale de la stratégie financière et économique, mais ce débat est aussi l'occasion de garder vivantes ses origines intellectuelles, de rappeler que la participation, « grande question du- XX -siècle c'est d'abord la sauvegarde de l'homme. Il s'agit bien d'« un idéal, un élan, un espoir » permettant à l'homme, « bien qu'il soit pris dans les engrenages de la pensée mécanique de voir « sa condition assurée » afin qu'il garde sa dignité et qu'« il exerce- enfin - ses responsabilités ». Je laisse maintenant la parole à mon collègue Dany Wattebled, qui va évoquer la question de l'actionnariat salarial.

assure une convergence des intérêts entre patronat et salariat. À l'heure de la réforme en profondeur de la gouvernance de l'entreprise, et à quelques jours des annonces du Président de la République, l'amélioration de ce type de dispositif est donc pleinement d'actualité. Le principe de cette participation des salariés à la vie de l'entreprise à travers un mécanisme d'actionnariat salarial n'est pourtant pas une idée nouvelle. Bien avant l'ordonnance gaullienne du 17 août 1967, la question de la participation financière des salariés au capital de l'entreprise avait été posée par une ordonnance du 7 janvier 1959. Cette ordonnance est le premier texte législatif instituant, en France, une formule de participation financière. Elle incarnait parfaitement cette alliance du capital et du travail souhaitée par le général de Gaulle. À partir des années soixante-dix, ce régime d'actionnariat salarial a connu une accélération par une série de lois plus ou moins complexes. Ces lois ont mûri l'idée d'une participation actionnariale des salariés, tout en nourrissant un système complexe et pesant. Les deux décennies suivantes ont d'ailleurs connu un véritable foisonnement de textes à ce sujet. Dans une actualité politique plus récente et dans un souci de simplification de ces mécanismes, la loi Macron du 6 août 2015 a cherché à redynamiser ce dispositif à travers deux mesures les attributions d'actions gratuites et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Il s'agit de revisiter le dispositif de l'actionnariat salarial avec des critères élargis et des méthodes remises à plat. Toutes ces initiatives législatives ont conduit notre pays à devenir le champion européen de l'actionnariat salarial. Ainsi, 76 % des entreprises françaises ont des plans d'actionnariat, contre une moyenne européenne de 36 % des salariés français sont actionnaires de leur entreprise, contre une moyenne de 22 % en Europe. Cette dynamique n'est pas seulement française ; elle s'observe également à l'échelle européenne. Aujourd'hui, sur 2 335 entreprises européennes représentant 99 % de la capitalisation boursière, un tiers placent les salariés en position stratégique ou déterminante dans le contrôle du capital de leur entreprise. Cette situation redonne donc le pouvoir aux salariés de participer directement à la gouvernance de l'entreprise. Elle leur permet aussi de se protéger contre la réorientation des activités entrepreneuriales ou une possible délocalisation vers un pays étranger.

Depuis des années, les précédents gouvernements ont privilégié des politiques de soutien à la consommation, plutôt que des incitations à l'actionnariat salarial et à l'épargne. La hausse du forfait social depuis 2012 est le témoin de ce choix du court terme plutôt que de l'avenir. Il faut revenir sur ces mesures. Cette situation invite en effet à la plus grande prudence quant à la pérennité de ces mécanismes. Si nous voulons simplifier les dispositifs de participation et tenir la promesse d'une revalorisation du travail des Français, alors des mesures énergiques doivent être rapidement prises à ce sujet. Tenons l'engagement de faire payer le travail, ajoutons une ligne supplémentaire au bulletin de paye de nos concitoyens récapitulant leur participation au capital des entreprises. Il faut qu'à la fin du mois le salarié puisse évaluer son effort au regard de son salaire, de ses cotisations sociales et de sa participation financière à l'entreprise. J'en viens à ma question, monsieur le secrétaire d'État. Le Président de la République a lancé un signal fort en évoquant la nécessité de repenser la participation financière des salariés à l'entreprise. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants souhaite savoir quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre pour défendre l'actionnariat salarial et lever les derniers freins

l'équité. Si l'on demande aux salariés d'accepter une plus grande part de risque dans un monde où les mutations économiques font qu'ils peuvent être soumis à des ruptures de carrière, et où la linéarité de l'exercice d'une profession dans un secteur d'activité ou dans une entreprise n'est plus la règle,

Cette part peut d'ailleurs être significative. En moyenne, elle s'élève autour de 2 500 euros par an, soit plus que l'équivalent d'un treizième mois pour de très nombreux salariés. Le deuxième enjeu, c'est

parce que l'épargne salariale, c'est un outil puissant pour le financement de l'économie, avec des encours qui s'élèvent aujourd'hui à 130 milliards d'euros, qui sont majoritairement investis en actions et qui viennent donc alimenter nos entreprises.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les dispositifs de participation et d'intéressement, enrichis ultérieurement par les outils d'épargne salariale, datent maintenant d'un demi-siècle. demi-siècle. Ils demeurent aujourd'hui un vecteur essentiel de justice sociale, en permettant l'affectation d'une partie des résultats des entreprises à un complément de rémunération pour les salariés. Ils sont aussi considérés comme un facteur important de motivation et contribuent à la compétitivité des entreprises. Si les sommes distribuées ou épargnées, qui représentaient 16,9 milliards d'euros en 2015, avec un montant moyen par salarié bénéficiaire de 2 422 euros, progressent de manière significative- de 5 % à 7 % entre 2014 et 2015 -, le nombre de salariés concernés a tendance, en valeur absolue ou en pourcentage, à stagner et même à diminuer.

d'une prime. Si la part de l'épargne salariale progresse, l'ensemble du dispositif semble s'essouffler. Cette situation est pour partie la conséquence de la très forte augmentation du forfait social : la contribution patronale est passée de 2 % en 2009 à 20 % en 2012, et ce malgré l'institution de taux dérogatoires pour certaines catégories dans la loi du 6 août 2015, dite loi Macron. Pour relancer ces dispositifs participatifs, il semblerait opportun de poursuivre les efforts engagés par la loi d'août 2015, en ramenant à un niveau moins dissuasif le montant du forfait social, en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement est-il prêt à s'engager dans cette voie ? La Madame la sénatrice, vous le savez, la mise en place de la participation n'est obligatoire qu'à partir de 50 salariés, mais les autres entreprises peuvent parfaitement le faire de manière facultative. Par ailleurs, les entreprises de toute taille peuvent négocier des accords d'intéressement. Aujourd'hui, 16,5 % des employés des entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'au moins un dispositif d'épargne salariale,

à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement dans les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent, pour la première fois- c'est le caractère incitatif de la mesure -, un accord de participation ou d'intéressement.

de moins de 50 salariés sont concernés. La volonté d'étendre cette « belle invention gaulliste », selon les termes mêmes du Président de la République, est un objectif louable. Ma question portera sur la méthode à employer. Le Gouvernement semble vouloir donner un caractère obligatoire au mécanisme de la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés, comme cela existe aujourd'hui pour celles qui sont au-dessus de ce seuil. Je ne pense pas qu'il faille privilégier cette voie coercitive.

Ensuite, il serait contradictoire de renforcer les contraintes des petites et moyennes entreprises, après avoir prôné leur allégement. Le calcul de la participation, qui est complexe, nécessite le concours d'un expert-comptable, ce que l'on ne peut pas exiger d'un petit entrepreneur. Enfin, cette piste entre en contradiction avec les conclusions du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié, le COPIESAS. En 2014, son vice-président, Christophe Castaner, remettait un rapport au précédent gouvernement, comprenant 31 propositions pour une réforme de l'épargne salariale. Il excluait précisément d'abaisser le seuil de 50 salariés, au-delà duquel la participation à l'épargne salariale est obligatoire.

en France, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est une forme d'intéressement. Cette participation permet la redistribution d'une partie des bénéfices réalisés. réalisés. Selon la dernière étude de la direction de la recherche du ministère du travail, environ 8 millions de salariés sont concernés par ce dispositif. En 2015, seulement 55 % des salariés du privé avaient accès au système d'intéressement, de participation et d'épargne salariale. Près de 16 milliards d'euros leur ont été versés. Le 15 octobre 2017, le chef de l'État a exprimé sa volonté d'améliorer cette belle invention gaulliste. Il souhaite lancer une grande réflexion sur l'entreprise, notamment en revisitant l'intéressement et la participation. La philosophie que porte le projet économique et social d'Emmanuel Macron est maintenant bien connue. Le Président de la République veut transformer en profondeur le monde du travail et les relations entre salariés, entreprises et partenaires sociaux. Sans attendre la future loi « entreprises », le Président a indiqué son cap. Je le cite : « L'entreprise, ça ne peut pas être simplement un rassemblement des actionnaires, notre code civil le définit comme cela. L'entreprise est un lieu, où des femmes et des hommes sont engagés. Certains mettent du capital, d'autres du travail. » le ministre de l'économie a expliqué que la participation, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, pourrait être étendue aux petites et moyennes entreprises. « C'est une question de justice, une entreprise ne tourne pas toute seule », a-t-il indiqué. Ma question est la suivante : pouvez-vous indiquer à la représentation nationale comment le Gouvernement pense mettre concrètement en oeuvre la volonté du Président de la République ? Quels seront les grands axes de ce chantier, notamment pour les entreprises les plus fragiles ?

je voudrais non pas élargir le sujet, mais le prendre dans toute sa dimension. À tous ceux qui veulent réaffirmer, à juste titre, la place des salariés dans l'entreprise et, comme l'a réaffirmé le porte-parole du Gouvernement, changer la gouvernance, nous répondons : Chiche ! Démocratisons les entreprises, les entreprises, accordons de nouveaux pouvoirs aux travailleurs ! En effet, le MEDEF et de nombreux patrons confondent allégrement l'entreprise et ses actionnaires, l'entreprise et son chef. l'entreprise, c'est avant tout l'ensemble des travailleurs qui la compose. Ce sont eux qui la font vivre, qui créent les richesses. À l'heure où l'exigence de démocratie est une aspiration largement partagée, l'entreprise reste largement une institution monarchique. Dès qu'il s'agit de l'entreprise, la démocratie est- malheureusement -un mot tabou. Il est donc temps de faire prévaloir d'autres choix que ceux qui ont été faits jusqu'à présent. Par exemple, plutôt que de fusionner les instances représentatives du personnel, créons des droits nouveaux d'intervention et de décision dans la gestion des entreprises pour les salariés et leurs représentants. Au lieu de réduire, comme l'ont fait les lois Macron et El Khomri, les pouvoirs du comité d'entreprise en cas de plan de sauvegarde de l'emploi, de licenciement et de restructuration économique, élargissons au contraire les droits d'intervention et de proposition des salariés et de leurs représentants. Pourquoi ne pas doter les comités d'entreprise d'un pouvoir effectif de contre-proposition économique ? Et dans certains domaines, qui touchent directement à la vie des salariés, tels que le plan de formation, le recours aux emplois précaires et à la sous-traitance, les heures supplémentaires ou le temps partiel,

est supérieur à 50 % des effectifs. On touche là une question de dignité du salarié, qui affecte directement son projet de vie. Plutôt que des mesures réglementaires, ne faudrait-il pas, pour régler ces questions, donner plus de pouvoirs aux représentants des salariés ? Qu'en pensez-vous ?

importante. La participation des salariés dans l'entreprise est reconnue de longue date en France. Des étapes ont été franchies et l'objectif général d'association des salariés à la création de valeur

Je veux que tous les salariés aient leur juste part quand les choses vont mieux. » Ce ne sont pas mes mots, mais ceux qui ont été prononcés par le Président de la République lors de son intervention télévisée du 15 octobre dernier. Il a souhaité rappeler la nécessité de partager les fruits de la réussite des entreprises avec les salariés, en développant des dispositifs de participation et d'intéressement. C'est un chemin vers lequel la majorité précédente, sous l'impulsion du président Hollande, s'était engagée en abaissant, par exemple, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le taux du forfait de 20 % à 8 % pendant les six premières années suivant la première mise en place d'un dispositif d'épargne salariale. Le porte-parole du Gouvernement, M. Castaner, a même prolongé la pensée du Président, en indiquant que l'objectif était de faire entrer les salariés au conseil d'administration des entreprises afin d'en transformer la gouvernance et d'améliorer le dialogue social. Mais, en même temps, le 18 octobre, le ministre de l'économie s'est montré, de son côté, très réservé sur ce point, en indiquant que l'octroi d'un pouvoir de décision aux salariés n'était pas une évidence. C'est à n'en plus savoir quelle est la ligne politique du Gouvernement ! S'agit-il de s'orienter vers un dispositif de codécision à l'allemande ou de louper, encore une fois, le coche de la modernisation des relations sociales en France ? Je n'ose pas croire que l'admiration de l'exécutif pour le modèle allemand ne porte que sur le pire et jamais sur le meilleur. Les salariés doivent avoir leur mot à dire sur les dispositifs de participation dans leur entreprise. Donner du pouvoir aux salariés dans les conseils d'administration, c'est répondre à un souci de justice et d'efficacité.

Vous l'avez rappelé, la philosophie du Président de la République est très simple- c'est la raison pour laquelle les Français l'ont élu : il faut que le travail paye et il faut qu'il paye mieux

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les débats de cet après-midi mettent en évidence l'importance d'apporter un regard neuf sur la question de la participation. Il faut repenser en profondeur les mécanismes d'intéressement et de l'actionnariat salarial pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Il faut aussi, et peut-être même surtout, en faire la publicité pour assurer leur développement rapide. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, il faut que le travail paye et, pour matérialiser cette réforme, que la participation financière soit effectivement visible dans le salaire mensuel de nos compatriotes. Cela pourrait faire l'objet d'une ligne supplémentaire sur le bulletin de paye, ainsi que nous l'évoquions plus tôt dans l'après-midi, en introduction de nos débats. Cette idée aurait, en outre, le mérite de changer le regard des Français sur leur paye mensuelle. La participation financière des salariés dans l'entreprise ne fait pas débat. Je crois que nous sommes tous favorables à ce que les employés aient une place consacrée au sein de l'entreprise et qu'ils soient capables de protéger leur activité contre les délocalisations ou les réorientations d'activité. Le bilan reste cependant en demi-teinte, comme je le disais précédemment. Aussi, nous devons redoubler d'efforts. Pour accompagner le développement de ces outils, il faut donc communiquer auprès des Français, les convaincre de la dimension positive de ces dispositifs de participation financière. Des actions de communication doivent ainsi être entreprises pour mieux faire connaître ces dispositifs. Cette politique tient sur deux jambes : d'un côté, un renforcement de l'usage de la participation financière par les entreprises ; de l'autre, une sensibilisation des employés à la pertinence de ces outils et à leur rôle de levier Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte donc sur la valorisation de la participation financière : quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer la communication autour de ces dispositifs ?

car, je suis d'accord avec vous, la question de l'identification, sur le bulletin de paie, de ce que représente la participation est un élément permettant à chaque salarié

et ont vocation à être pérennisées. En 2017 s'est tenue la première édition de la semaine de l'épargne salariale. Ce n'est pas faire injure à cet événement que d'avouer qu'il

Nous sommes très ouverts pour conduire une campagne de communication offensive, différente à la fois dans le message, dans la manière de le porter et dans le support pour le diffuser. Toute idée innovante et disruptive est évidemment la bienvenue sur ce sujet.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question porte sur un thème cher à notre président de séance, Jean-Marc Gabouty. L'accès des salariés aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale est directement lié à la taille des entreprises. En effet, ceux-ci sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés et demeurent facultatifs dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans les PME et TPE de moins de 50 salariés, seuls 16,5 % des salariés sont couverts par ces dispositifs et cette proportion a tendance à s'effriter. Sur la totalité des sommes distribuées ou épargnées, les salariés de cette catégorie d'entreprises ne reçoivent qu'environ 500 millions sur un total de 16,9 milliards d'euros.

des mesures plus incitatives en diminuant le niveau du forfait social ou en le rendant progressif. Les entreprises de cette catégorie qui mettraient en place pour la première fois, et volontairement, un régime de participation ou d'intéressement pourraient être exonérées du forfait social pendant les trois premières années, puis bénéficier d'un taux de 8 % les trois années suivantes, enfin de 16 % au-delà. Monsieur le secrétaire d'État, quelles mesures le Gouvernement peut-il envisager pour permettre à un plus grand nombre de pour permettre à un plus grand nombre de salariés des PME et TPE d'avoir accès au régime de participation, d'intéressement et d'épargne salariale

d'entrer dans le dispositif. Nous sommes prêts, dans le cadre du groupe de travail et du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, dans lequel nous sommes engagés avec Bruno Le Maire, à réfléchir de nouveau à ces sujets, qu'il faut néanmoins manier avec précaution

Pourquoi ne pas plutôt revoir la taxation trop élevée de ce dispositif, principal obstacle à son développement ? Ma question portera donc sur le forfait social. Je rappelle que cette taxe est passée de 2 % en 2009 à 8 % en 2011, avant de faire un bond à 20 % en 2012, sous la présidence de François Hollande, décourageant les employeurs d'utiliser ce mode de rémunération complémentaire. Avec la loi du 6 août 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait prévu le retour à un forfait social réduit à 8 mais uniquement pour les TPE et PME volontaires entrant pour la première fois dans le dispositif, et ce durant 6 ans. Pourquoi ne pas avoir été plus loin en exonérant totalement du forfait toutes les entreprises de moins de 50 salariés ? De plus, il a été créé une discrimination entre les sociétés ayant déjà signé un accord avant 2011 et celles qui l'on fait après 2011. Monsieur le secrétaire d'État, si vous voulez donner de la liberté aux entreprises, si vous voulez développer l'épargne salariale, alors, chiche, allez jusqu'au bout : enlevez le forfait social pour toutes les entreprises des travailleurs indépendants, dont la rémunération est leur résultat net, allez-vous déterminer vous-même cette rémunération en ponctionnant sur le résultat une part réservée à la participation ? Je vous remercie de bien

Je crois à la liberté de l'entrepreneur, qu'il soit grand ou petit, d'organiser au sein de l'entreprise, avec les salariés et ses collaborateurs, la manière dont on peut répartir les fruits du travail les bénéfices engendrés. Nous y sommes très attachés. En tout cas, c'est dans cet esprit que travailleront les deux rapporteurs sur ce sujet important de la participation et de l'intéressement. Il n'est pas question d'obliger nous croyons à la formule incitative. Vous soulignez l'apport de la loi du 6 août 2015, et il faut effectivement se féliciter de la baisse du forfait de 20 % à 8 %, laquelle a permis à des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne d'entrer dans le dispositif.

l'attaque sur les dépenses publiques est importante et où nous cherchons à faire des économies pour permettre de retrouver une trajectoire financière plus pérenne, en tout cas plus soutenable, compte tenu des engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires. C'est toujours en respectant cette que se joueront les discussions sur le sujet, sachant que les dispositifs d'épargne salariale ne s'adressent pas aux indépendants, qui recueillent, eux, directement le bénéfice de leur travail à travers la valorisation de leur propre

lorsqu'elles réalisent un bénéfice suffisant. Elle est un outil de partage des bénéfices, mais aussi d'épargne, qui bénéficie d'avantages fiscaux. Le Président de la République a récemment annoncé un vaste chantier sur l'entreprise et un dialogue social redéfini, redéfini, afin que tous les salariés puissent recevoir les fruits des bons résultats de l'entreprise. En effet, seuls 56 % des salariés du privé bénéficient des outils de la participation, de l'intéressement

83 % des salariés ont accès à au moins une formule d'épargne salariale, le chiffre tombe à 20 % dans les entreprises de 10 salariés et à 12 % dans les entreprises de moins de 10 salariés. Nous connaissons les freins à ce développement : complexité de gestion des dispositifs, préférence donnée aux primes et, surtout, illisibilité des dispositions fiscales, qui sont imprévisibles. Rendre le dispositif de participation obligatoire sans prendre en compte ces spécificités me paraît dangereux pour toutes ces petites entreprises qui ont le souci de développer leur activité, et

doit se concentrer sur son activité avant de se concentrer sur l'encadrement réglementaire, législatif, comptable de son activité. En effet, s'il consacre son temps à autre chose qu'à son activité, je crains qu'il ne la développe pas.

c'est-à-dire en partant des expériences vécues. C'est aussi l'objet des auditions de ces groupes de travail. Certes, nous auditionnerons les traditionnels corps constitués, mais nous auditionnerons aussi ceux, qui, bien souvent, ne se sentent pas représentés, ont eu des parcours entrepreneuriaux qui les ont tenus à l'écart des instances délibératives

permettrait de faire profiter les salariés des richesses créées par leur entreprise. Je voudrais m'associer à mon collègue Dominique Watrin pour regretter que l'on n'ait pas pu parler de la participation comme droit démocratique nouveau accordé aux salariés. Je voudrais également soulever un paradoxe aujourd'hui, le choix de cette participation justifie ou occulte pour une part le refus des employeurs de revaloriser les salaires de manière importante, tout comme, d'ailleurs, celui de l'État d'augmenter le montant du point d'indice pour les fonctionnaires. Si la rémunération des salariés augmente par le truchement des primes liées à la participation aux résultats des entreprises, il n'est pas inutile de préciser qu'elles sont exemptes de cotisations sociales. À l'heure des saignées budgétaires dans le domaine de la santé, singulièrement au détriment des hôpitaux, on peut s'interroger sur cette exonération des entreprises concernant le financement de la sécurité sociale, d'autant que, contrairement aux salaires, les sommes versées au titre de la participation ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la retraite des salariés. En réalité, la participation est une rémunération aléatoire, discrétionnaire, dont les résultats dépendent du bon vouloir des dirigeants des entreprises. Par exemple, alors que les salariés participent au quotidien à la production des richesses, leurs salaires ne vont augmenter que de 1,8 % en 2017, tandis que les entreprises du CAC 40 ont réalisé 50 milliards d'euros de bénéfices au premier semestre 2017, soit une hausse de 24 % par rapport à 2016.

déjà évoquée tout à l'heure, de la révision de la formule du calcul de la participation pour en faire un instrument plus juste et plus équitable de répartition des fruits du résultat de l'entreprise. À la fin, quand l'entreprise est bénéficiaire, qu'elle a des résultats importants, c'est grâce à la totalité des personnes qui la composent. Nous Nous sommes ouverts à une réflexion qui permettrait une répartition plus juste entre les différentes échelles de la grille

travailler à y remédier, de manière sereine, sans opposer le monde de la fonction publique et celui du salariat. Enfin, ouvrir la question de la participation et de l'intéressement dans la fonction publique est aussi, sans doute, un moyen de la faire évoluer,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la participation dans une entreprise peut avoir plusieurs origines. Elle peut parallèlement atteindre plusieurs objectifs. Il existe un véritable problème dans notre pays : la transmission des entreprises. Quand on est chef d'entreprise et que l'on veut transmettre son entreprise pour cause de départ à la retraite ou pour raisons personnelles, cela relève parfois du parcours du combattant. Dans certains cas, un ou plusieurs salariés, ou même un tiers, seraient intéressés pour reprendre une entreprise à laquelle ils sont très attachés.

Or ce dispositif d'incitation manque dans notre législation. Ce mécanisme pourrait être une solution de reprise des entreprises par des acteurs qui limiteraient le risque de défaillance. Cette solution pourrait être élargie à des tiers à l'entreprise. Le rachat progressif des capitaux par la participation dans le capital favoriserait l'entrée dans l'entreprise d'un repreneur qui augmenterait ses parts peu à peu. Dans nos zones rurales, la transmission d'entreprise est difficile parce que les repreneurs locaux ne sont pas si nombreux. Alors, cette participation pourrait favoriser les acteurs locaux et limiter ainsi les risques de délocalisation et de fermeture.

qui souhaitent apporter leur épargne dans le tissu économique local. C'est certainement un concept à imaginer ou à réimaginer. Vous comprenez, monsieur le secrétaire d'État, que cette question de la transmission d'entreprise me tient particulièrement à coeur. coeur. Il est toujours cruel de voir les entreprises de son territoire fermer ou partir, alors que des personnes locales auraient pu reprendre si l'on avait su anticiper cette cession. J'espère que vous tiendrez compte de cette contribution dans votre prochaine réflexion concernant la participation dans les entreprises. La parole

est intervenue en 2006. On n'est donc pas vraiment dans la PME de nos territoires, ni dans des enjeux très locaux. Néanmoins, ce mécanisme existe. Il est extrêmement contraignant- je vous fais grâce des différents éléments nécessaires pour sa mise en oeuvre. Pour autant, c'est un dispositif intéressant dans le cas d'une reprise : jusqu'à 95 % de l'actif peut-être investi en titres de l'entreprise et la poche d'actifs liquides peut-être réduite à 5 % de la valeur de l'actif du fonds

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Président de la République a annoncé une grande discussion sur la « philosophie de l'entreprise ». Ma question portera sur l'étendue de la réforme envisagée. Comme nous venons de l'évoquer, il s'agirait tout d'abord de renforcer les mécanismes d'épargne salariale, « belle invention gaulliste », selon l'expression présidentielle, afin de mieux associer les salariés aux résultats de leur entreprise. Mais il semble que le Gouvernement souhaiterait également associer davantage les salariés à la gestion de l'entreprise en modifiant la composition des instances de gouvernance. Il s'agit d'un sujet récurrent. Deux lois ont été adoptées sous le gouvernement précédent. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a imposé la présence d'un ou plusieurs administrateurs salariés dans les entreprises d'au moins 10 000 salariés ayant leur siège social à l'étranger, et à partir de 5 000 salariés en France. Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les seuils sont passés respectivement à 5 000 et 1 000 salariés. Encore plus récemment, le projet de loi visant à autoriser le Gouvernement prévoyait une « amélioration des conditions de représentation et de participation » des salariés pour « un effectif dépassant un certain seuil », ce qui laissait augurer une nouvelle baisse des seuils. En CMP, le Sénat a obtenu la mention de l'impossibilité de revenir sur les seuils actuels afin d'éviter l'instabilité législative qui en découlerait, ainsi que de nouvelles contraintes pour les entreprises. Finalement, le Gouvernement a abandonné son projet aucune mention de la participation des salariés aux conseils d'administration ne figure dans les ordonnances. Cependant, le Président de la République semble souhaiter introduire de nouveau ce sujet dans une loi sur la transformation des entreprises, qui serait présentée au printemps 2018. Il faudrait que les intentions du Gouvernement en la matière soient plus claires, car il est inutile d'envoyer sans cesse des signaux négatifs aux investisseurs. Pourriez-vous nous préciser ce que souhaite faire le Gouvernement à ce sujet, monsieur

ce qui implique de l'écoute, des échanges. Nous attendons de nous faire un peu bousculer sur ces sujets. Comme le Président de la République l'a dit dans son intervention télévisée du 15 octobre, il faut mieux répartir les fruits et les bénéfices des entreprises. Si une entreprise va bien, les salariés doivent pouvoir en bénéficier plus largement, quand aujourd'hui seulement un salarié sur deux bénéficie des mécanismes de participation ou d'intéressement. C'est donc bien l'objectif qu'auront Agnès Touraine lorsqu'ils détermineront la manière dont ils vont conduire ces travaux. La question de la gouvernance et de la participation des salariés aux organes de direction des entreprises est un sujet qui peut être ouvert dans le cadre de ce groupe de travail.

peut-être pouvons-nous envisager un échange dans le cadre de ces groupes et des propositions qui seront formulées et livrées à la consultation publique début janvier, avant d'engager le processus législatif plus traditionnel de construction avec les différents services. Sachez-le, si la participation devait s'étendre, il faudrait qu'elle soit adaptée à la spécificité de chacune des entreprises. Je le répète, il est question non pas de faire une loi pour chaque type d'entreprise, mais de trouver au plus près de la situation, des réalités de chacune des entreprises et de chacun des secteurs concernés le meilleur moyen d'associer les salariés aux fruits et aux bénéfices réalisés par les entreprises.

comme cela a déjà été souligné, les signes de croissance pour notre pays s'améliorent cette année, avec des perspectives favorables pour l'avenir. Nous ne pouvons que nous en réjouir, et notre rôle de responsables politiques est bien d'accompagner ce mouvement positif et, surtout, de ne pas l'entraver. Pour ce faire, deux leviers sont pointés pour la relance de notre économie : favoriser la consommation en augmentant le pouvoir d'achat des Français et réinciter les Français à investir dans leurs entreprises pour créer de la richesse sur notre territoire. L'annonce du Président de la République de développer la participation dans les entreprises accompagne ce mouvement. La réforme proposée pourrait passer par de nouvelles dispositions, des exonérations fiscales et sociales, pour autant, veillons-y, rigidifier le dispositif existant, notamment pour les petites entreprises. Profiter de développer la participation pour favoriser l'accès des salariés au capital des entreprises serait un signe positif afin, d'une part, valoriser leur travail et, d'autre part, de recréer du lien, de la communauté d'intérêts entre le salarié et la structure pour laquelle il travaille.

plus généralement, par d'autres acteurs privés et associés d'un même territoire, afin de renforcer la notion de coopération et de solidarité de territoire. Augmenter le capital, c'est redonner à l'entreprise une capacité d'investir, c'est favoriser sa recherche et développement pour mieux se projeter sur de nouveaux marchés.

de ne pas confondre l'accès au capital d'une entreprise par l'augmentation de ses fonds propres avec ce qui ne pourrait être, sans cette augmentation de capital, que de simples transactions spéculatives sur des opérations d'achat-vente de parts sociales existantes. Ce dernier cas ne favoriserait que la rente, et non pas le développement ou la croissance de l'entreprise.

Madame la sénatrice, il n'est évidemment pas question au travers de ce projet de loi d'encourager un quelconque phénomène de spéculation,

ce phénomène que nous souhaitons amplifier, en favorisant l'investissement des Français dans notre économie, dans nos entreprises, plutôt qu'ailleurs.

-de reflécher, de réorienter le capital productif vers nos entreprises et vers le financement de nos entreprises. Pour ce faire, l'une des pistes consiste à identifier des investissements qui donnent du sens, d'éviter les phénomènes spéculatifs ; c'est ce que l'on appelle « les investissements socialement responsables ». Ce sont des mécanismes que l'on retrouve dans les entreprises où la France a d'ailleurs une vraie signature à l'étranger, avec des entreprises qui connaissent de grands succès. Je pense, par exemple, à KissKissBankBank, qui vient de nouer un partenariat avec une entreprise bien connue de nos concitoyens, une grande banque française, la Banque Postale. Il y a là des éléments intéressants en termes d'investissements socialement responsables. Notre vision est, me semble-t-il, partagée : c'est celle d'une France où les Français sont incités à prendre des risques, à orienter leur épargne plutôt vers les entreprises françaises qu'ailleurs,

en termes d'image pour le modèle financier. Pour ce qui me concerne, je ne fais pas partie des ennemis de la finance. Je pense que la finance est au service de l'entreprise, de l'économie réelle et des emplois. Le pire service à lui rendre est de l'autoriser à faire n'importe quoi, ce qui ne sera pas le cas dans ce cadre de ce projet.

C'est le constat qu'une grande partie de la classe politique et des experts en tout genre tire depuis de nombreuses années, sans trop savoir comment régler cette épineuse question et engager un profond changement des mentalités. Ce débat n'est pas purement technique. Il est tout aussi philosophique, ce qui lui donne un caractère particulièrement complexe. Le Président de la République, lors de son entretien télévisé, a laissé entendre qu'il comptait ouvrir un nouveau chapitre de la participation dans l'entreprise. Sans en préciser la philosophie, il a néanmoins insisté sur la nécessité d'intégrer plus et mieux les salariés à la vie de l'entreprise. Je le rejoins sur ce point et partage la volonté d'engager une indispensable évolution de l'entreprise : le regard qu'elle porte sur ses salariés et la manière dont elle doit les associer à sa réussite. Peut-on et doit-on aller plus loin ? Je le crois. Ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus que de créer un simple mécanisme à l'endroit des salariés, c'est définir une nouvelle relation dans l'entreprise : une relation de confiance, de respect mutuel, d'évolution commune et de réussite partagée. L'investissement de tous, à des degrés divers, doit être récompensé. Encourager la participation, c'est mieux associer les salariés de l'entreprise aux réussites et aux échecs ; c'est les sensibiliser, au-delà de leur carrière, aux enjeux globaux de l'entreprise, aux enjeux du marché sur lequel elles évoluent, aux perspectives d'avenir et de développement. Toutes ces questions sont complexes. Elles méritent un véritable débat, apaisé et dépassionné pour tenter d'apporter des réponses aux Français qui attendent une meilleure redistribution et un meilleur partage de la réussite. Il est temps de montrer que les entreprises ne servent pas exclusivement des intérêts particuliers et qu'elles contribuent à la réussite économique de tout un pays. Et je crois que ce principe doit être inscrit dans la loi. Aussi, que compte faire le Gouvernement, de manière très concrète, pour développer la participation au sein de l'entreprise ? La parole monsieur le ministre,

au début de mon propos. En effet, si l'on considère que la relation dans l'entreprise ne peut se construire, s'imaginer ou se penser que dans le cadre de très grandes entreprises avec des logiques très verticales puisque les personnes ne se connaissent pas forcément-

salariés. L'association directe des salariés à l'entreprise est porteuse de réussite et favorise la compétitivité des entreprises, comme cela a été dit à de nombreuses reprises. Néanmoins, j'aimerais insister sur deux points. Premier point : la nécessaire simplification des dispositifs de participation et d'intéressement, notamment pour les TPE et les PME. Je suis certaine que le Premier ministre tiendra ses engagements en matière de réduction des normes. Mais le souci de pragmatisme du Gouvernement doit se traduire surtout et avant tout par plus de lisibilité dans les dispositifs. En effet, les freins techniques et juridiques sont encore trop nombreux, singulièrement pour les petites entreprises. Deuxième point : la stabilité de la fiscalité applicable à la participation. Entre sa création en 2009 et aujourd'hui, le taux du forfait social unique n'a fait qu'augmenter, passant de 2 % à 20 %, ce qui entraîne une véritable frilosité de la part des entreprises. de la sécurité sociale pour 2018 est consacré à l'augmentation du pouvoir d'achat des actifs, le Gouvernement souhaite supprimer le mécanisme des « taux historiques » des prélèvements sociaux pour les gains acquis à compter du 1 janvier prochain. cette mesure législative, on inscrit dans le marbre une instabilité fiscale qui fragilise les mécanismes de participation. Ma question est simple : pourquoi adopter une telle mesure, qui brouille les messages adressés aux employeurs et aux salariés, alors que des projets phares de la réforme de la participation sont en cours, notamment avec la grande concertation que vous organisez ? Comment voulez-vous favoriser une épargne longue pour soutenir l'investissement, en particulier dans les PME et les TPE ?

Tout ce que l'on peut faire pour avoir des lois moins bavardes, des textes plus clairs, une réglementation plus compréhensible pour nos citoyens et les entreprises

Dans mon portefeuille, j'ai la responsabilité de l'attractivité financière de la Place de Paris. Lorsque je vais à l'étranger- je me rendrai tout à l'heure à l'Élysée où le Président de la République reçoit de très nombreux investisseurs étrangers prêts à venir voir ou, en tout cas, à regarder avec un oeil attentif ce que nous portons -, la question de la stabilité fiscale et sociale de nos mécanismes est assez centrale.

fondamental concernant la « participation dans l'entreprise, outil de croissance et perspectives ». C'est un thème particulièrement important pour l'emploi et l'activité économique. Nous le vivons au quotidien dans nos départements respectifs, nous sommes toutes et tous attachés à l'activité économique sous toutes les formes, en particulier dans le monde rural, qu'il convient aussi de soutenir.

lien de confiance, leur travail, leur implication, leurs motivations constituent le rattachement à l'outil de travail et à la réussite. C'est un combat permanent, où tous ont un rôle à jouer. Cependant, il existe des limites, des embûches. Les chefs d'entreprise s'ouvrent souvent à nous au sujet de la complexité dans les démarches : code du travail, sécurité, bien-être au travail, difficultés à recruter, à embaucher, charges sociales et fiscales, concurrence déloyale, complexité

est un compliment. Je ne sais pas si je finirai par être plus parisien que je ne suis bourguignon ... Ayant passé la moitié de ma vie en Bourgogne et l'autre à Paris, je suis sans doute à mi-chemin.

des hauts fonctionnaires des différentes directions de nos administrations respectives, des parlementaires et des corps constitués. Nous allons partir du réel, de cas très concrets de simplification, d'embûches administratives, d'embûches bancaires, de difficultés à avoir des relais de croissance, en vue de trouver des solutions très concrètes. Je le redis, je ne crois pas que la loi règle tous les problèmes. Je suis même intimement convaincu que certains problèmes peuvent être levés très rapidement par des petits verrous réglementaires, parfois même en engageant une action publique plus intelligemment concentrée sur certains éléments. C'est dans cet esprit que nous abordons le travail que nous venons d'engager sur ce projet important

de ce débat. C'est un moment important parce que nous sommes au début d'un travail de réflexion. Les différentes questions qui ont été abordées viennent teinter la manière dont on va travailler. Je vous invite le plus sincèrement du monde à apporter votre contribution, vos idées, votre expertise des territoires. Je ne veux pas que l'on nous explique que c'est un truc de start-uppers parisiens, car ce n'est pas le cas.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat que nous organisons ce soir à la demande de la commission

le parent pauvre des politiques publiques. Cette situation a des conséquences qui se répercutent, nous le voyons bien, lors des différents scrutins politiques. Le constat que nous avons fait est clair : la fracture territoriale s'amplifie ; la croissance des métropoles, qui étaient censées irriguer l'ensemble du territoire, a plutôt un effet d'appauvrissement des zones les plus fragiles ; de nombreux territoires, qu'ils soient ruraux, urbains ou périurbains, connaissent un recul, en termes d'activité, d'emploi, de services publics et de dynamisme Nous regrettons que, face à cette situation, l'État soit plus un spectateur qu'un acteur. Il nous paraît donc urgent de refonder la politique de l'aménagement du territoire.

Si nous considérons que le principal acteur en matière d'aménagement du territoire doit être le binôme région-EPCI, il n'en demeure pas moins que nous pensons indispensable que l'État redevienne stratège,

Nous souhaitons également- et je regarde spontanément Rémy Pointereau -que l'on avance dans la simplification des normes, comme le demande notre collègue. Par ailleurs, la politique d'aménagement du territoire doit essentiellement être basée sur la contractualisation. En outre, il nous paraît nécessaire que les dotations et subventions aux collectivités territoriales soient plus transparentes et équitables, et qu'elles comportent un aspect incitatif au regard de l'aménagement du territoire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme vient de le dire parfaitement le président Maurey, au fil des années, l'aménagement du territoire est devenu le « parent pauvre » des politiques publiques. Malgré le constat objectif d'une disparition progressive des services publics, notamment dans le monde rural, malgré le sentiment d'abandon d'un nombre important de nos concitoyens et malgré le cri d'alarme des élus locaux, rien- ou presque rien -ne change, monsieur le ministre Hervé Maurey vous a fait part des grands axes de propositions de notre groupe de travail. Depuis des années, et quels que soient les gouvernements concernés, nos territoires fragiles ont été oubliés. Il est donc grand temps de s'emparer pleinement de ces propositions et d'agir Je vais prendre un premier exemple : celui de la désertification médicale. C'est une réalité désormais bien connue, durement subie par une part toujours croissante de la population de notre pays- plus de 5 millions d'habitants vivent dans ces zones. Or, que font les pouvoirs publics pour y remédier ? Des plans ! Les mêmes plans depuis quinze ans ! C'est-à-dire un ensemble de mesures d'affichage ou à caractère incitatif qui ont fait la preuve de leur inefficacité et qui, aujourd'hui, ne sont clairement plus à la hauteur des enjeux. Nous sommes persuadés, au sein de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qu'il faut franchir une nouvelle étape et mettre en place une régulation de l'installation des médecins, comme cela existe pour les autres professions de santé. Cette mesure a été adoptée à plusieurs reprises par notre commission, mais a toujours été écartée des textes législatifs définitifs, alors qu'il s'agit d'une attente très forte des populations. Or il y a urgence. Il faut de vraies mesures. Deuxième exemple : la couverture mobile et numérique du territoire. Des objectifs ambitieux ont été fixés et réaffirmés voilà à peine un mois il s'agit, d'une part, du déploiement du « bon haut débit pour tous » dès 2020, d'autre part, d'« une disponibilité généralisée de la 4G », toujours d'ici à 2020. Mais que mettez-vous précisément, monsieur le ministre, derrière ces slogans, il est vrai séduisants ? Et quels sont les moyens que vous avez prévu d'y consacrer ? Nous étions déjà inquiets sur le respect des objectifs fixés pour 2022 ; comment allez-vous parvenir à les avancer, du moins pour partie, à 2020 ? Troisième exemple : le développement des infrastructures. Que ce soit pour l'entretien des infrastructures existantes ou pour les projets de nouvelles infrastructures, il est grand temps, selon nous, que le critère de l'aménagement du territoire prenne le pas sur celui de la rentabilité économique. Il n'est plus possible de tout analyser sous le seul prisme de l'intérêt économique à plus ou moins court terme. Ce calcul est de plus un mauvais calcul, car les choix que nous évitons ou reportons deviendront un jour ou l'autre nécessaires et infiniment plus coûteux. Monsieur le ministre, nos préconisations ne sont clairement pas entendues pour l'instant. Or, je le redis, aux yeux de tous les membres du groupe de travail de notre commission, la prise en compte de l'aménagement du territoire dans l'ensemble des politiques publiques est une priorité qui ne peut plus attendre. Pourriez-vous donc nous donner quelques éléments de nature à nous rassurer ? En effet, au-delà de nos propres interrogations, l'aménagement du territoire, l'égalité des territoires, la cohésion des territoires- peu importe comment on l'appelle, les problèmes se posent toujours dans les mêmes termes -, est bien le souci majeur des élus locaux et de nombre de nos concitoyens présents sur les territoires que nous représentons. La parole

ici, du haut de cette tribune, dont j'ai un peu l'habitude. J'ai écouté avec intérêt mes anciens collègues,

une politique d'aménagement du territoire de nature à réparer les nombreuses fractures donc vous avez relevé l'existence. Je vous remercie

point, par exemple, que les régions- et elles se lancent -ne s'occupent pas de l'aménagement de leur territoire. Et je sais qu'elles en ont bien la volonté. Les dynamiques territoriales ne se réduisent pas à l'image simpliste, trop souvent relayée, qui conduit à opposer les territoires les uns aux autres. Je n'utilise jamais l'opposition urbain-rural, parce que la situation des territoires est très différente à l'intérieur

Dans votre rapport, vous citez le géographe Roger Brunet, pour qui nous serions passés d'un territoire « à aménager » à un territoire « à ménager ». Le mot est d'ailleurs intéressant.

Vous avez raison de souligner « qu'il n'est plus possible, aux niveaux démographique et géographique, de considérer l'urbain et le rural comme deux entités bien définies qui s'opposeraient l'une à l'autre ». Nous sommes totalement d'accord. Les Les visions sur la « France périphérique » sont une grille de lecture. Des éléments de constat nécessitent une action. Bien sûr, je sais qu'il ne faut pas être trop schématique,

Je ne reviens pas sur le rapport de France Stratégie, que nous avons tous lu et relu, et, pour beaucoup d'entre nous, critiqué. France des métropoles serait la gagnante égoïste de la mondialisation et la France périphérique aurait tout perdu et n'aurait pas d'avenir. Or il est essentiel que cette France-là ait un avenir et que nous le construisions ensemble. Nous devons aussi nous garder de cette vision théorique qui résumerait notre pays à des espaces dynamiques, en reléguant une partie du territoire au rang de zones interstitielles- mot que je n'aime pas du tout. Représentant d'un territoire

en distinguant la campagne des villes, du littoral et des vallées urbanisées, où vivent 16 millions d'habitants dans plus de 10 000 communes. Si l'on ne peut construire une politique de cohésion du territoire sur l'opposition entre les territoires favorisés et les autres, il ne s'agit pourtant pas de nier- ce que je ne ferai pas -que certains territoires connaissent des difficultés considérables, qui se sont aggravées ces

Beaucoup a été fait pour les quartiers prioritaires, mais beaucoup reste à faire : le taux de chômage y est deux fois et demie supérieur à la moyenne nationale, le taux de pauvreté, deux à trois fois supérieur. Je pense aussi à certains centres-bourgs et à certains centres de villes moyennes dévitalisés, qui sont aujourd'hui un enjeu considérable parce que si nous n'intervenons pas rapidement, ces villes moyennes- même si elles ne sont pas toutes, heureusement, dans cette situation-là -connaîtront des difficultés encore plus importantes, avec la fermeture de commerces, l'absence d'emplois ou de formations, la dégradation du bâti, enjeu important. Dans les territoires peu denses, l'accès aux services est un problème primordial. Je connais les difficultés très concrètes liées à la fermeture progressive des services publics-

C'est un constat, et face à cela, il nous faut agir. Je veux revenir ici sur certains axes concrets d'intervention avant de partager avec vous ma vision de la méthode d'ensemble dont j'ai la charge comme ministre

Je suis aussi attaché à ce que l'État se préoccupe de l'accessibilité de certains territoires enclavés, que je connais peut-être mieux que d'autres pour subir cet enclavement plus que d'autres. Et s'il a été annoncé qu'on mettrait un frein à certaines grandes opérations, à grande vitesse, il est nécessaire d'entretenir nos routes nationales, il est nécessaire d'entretenir certaines voies ferrées qualifiées de « secondaires », car beaucoup de travaux n'ont pas été réalisés depuis longtemps. nécessaire aussi de lutter pour le maintien des services publics. Nous avons pris la décision d'accélérer le déploiement des maisons de services au public,

Vous avez parlé des déserts médicaux. Nous avons souvent échangé sur ce point dans cet hémicycle.

sur cette réalité-là. Une des priorités de notre action, c'est le déploiement du numérique. Vous y avez insisté dans votre rapport : c'est essentiel pour réparer les fractures territoriales. Parce que nous ne pouvons pas prendre le risque, ni les uns ni les autres, d'aggraver la fracture territoriale numérique, nous avons pris la décision d'avoir comme objectif le bon débit pour tous d'ici à 2020, le très haut débit d'ici à 2022. J'ai réuni à deux reprises au ministère les opérateurs, leur demander de prendre des engagements contraignants, conformément à la dernière loi Montagne. Les discussions sont toujours en cours, mais je suis assez optimiste au regard des réponses qui commencent à nous être faites. faites. C'est comme cela qu'on pourra avancer. Vous le savez aussi, l'État, dans son rôle d'État stratège auquel vous tenez, dispose de quelques moyens de négociation avec les opérateurs, et ces moyens seront utilisés si nécessaire. Il est indispensable d'accélérer la couverture numérique par l'installation en particulier de plusieurs milliers de pylônes supplémentaires pour avoir le bon débit- la 4G d'ici à 2020 -, mais aussi d'utiliser des technologies alternatives, que ce soit la montée en débit, la 4G fixe, le satellite. Je l'ai dit, nous avons une position claire et ferme vis-à-vis des opérateurs, avec aussi la protection des réseaux d'initiative publique portés par les collectivités et qu'il ne faut pas mettre en danger. Voilà des réponses précises à des questions précises. Bien sûr, nous ne savons pas encore quels seront tous les impacts de cette révolution numérique sur nos territoires, mais ils seront considérables et ils vont s'amplifier. En particulier, en matière de domotique ou en matière de nouvelles mobilités, les choses vont avancer considérablement dans les quelques années qui viennent et beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Il est normal d'aborder la question du volontarisme politique lorsqu'on évoque l'aménagement du territoire.

une période d'aménagement du territoire et de planification, qui ont été poursuivis dans les premières années de la V République, mais qui petit à petit, malheureusement, ont été abandonnés. Nous considérons aussi que les réformes territoriales ont entraîné un certain nombre de bouleversements. Je ne reviendrai pas sur la fusion des régions, sur ce que nous avons vécu.

heureuses. Sans vouloir faire un aparté, je pense que la situation actuelle n'est pas forcément la meilleure à laquelle il aurait été possible d'aboutir, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. ! Je n'oublie pas le rôle d'aménageur du territoire de certaines collectivités- j'ai parlé des régions. Le Président de la République a annoncé, ici au Sénat, le 17 juillet dernier, une pause dans ces réformes institutionnelles et que l'heure n'était plus au lancement de grands programmes publics d'aménagement. Je note, pour m'en réjouir, que votre rapport exprime des réserves sur le rôle de facilitateur de l'État, parce que ce rôle est venu remplacer celui d'organisateur. Ces craintes sont compréhensibles, mais tout de même, il vaut mieux que l'État soit facilitateur qu'empêcheur de conduire des projets sur les territoires ! Chaque fois que nous nous exprimons en particulier devant les services déconcentrés de l'État, le message que je transmets,

deux points. La politique contractuelle est indispensable. Néanmoins, nous sommes en train de faire le bilan des différents contrats qui existent entre l'État et les collectivités. Nous en sommes à plus de 1 100 contrats différents, le ministère de la culture semblant même être en première position. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut de la contractualisation, mais qu'il faut la simplifier pour y voir clair. Parce que la multiplication de centaines et de centaines- plus de 1 -de types de contrat n'est quand même pas un très bon exemple. Contrats de plan, contrats de ruralité, demain contrats de ville moyenne : nous allons poursuivre cette politique de contractualisation, mais en essayant de la simplifier,

Le Président de la République y déclarait : « Vous l'avez compris, je souhaite accompagner, encourager les initiatives, supprimer les verrous encore trop nombreux qui contraignent les territoires dans leur souhait de s'organiser mieux, en vue d'une action publique plus efficace. Cette liberté sera laissée aux élus locaux, en lien avec les représentants de l'État aussi, pour expérimenter de nouvelles politiques publiques, de nouvelles organisations des services publics, mais aussi pour innover en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et pour définir notre territoire de demain. aménagement du territoire », tout est dit ! Voilà sans conteste, monsieur le ministre, des propos qui donnent le tempo pour un nouvel âge de la politique d'aménagement du territoire et pour le fameux droit d'expérimentation.

À cette occasion, Mme la ministre Jacqueline Gourault est revenue sur le droit à l'expérimentation, aujourd'hui trop peu utilisé par les collectivités. Elle a rappelé, répondant en cela à l'engagement du Président de la République, combien il était nécessaire de le simplifier, alors même qu'il existe aujourd'hui l'obligation d'une généralisation de ces expérimentations sur tout le territoire au bout de deux ans ou d'un arrêt pur et simple. Pouvez-vous nous en dire plus, monsieur le ministre, sur les intentions du Gouvernement en la matière et peut-on imaginer que ce droit à l'expérimentation simplifié se transforme, à terme, en droit à la différenciation de l'action publique au regard des spécificités de nos territoires ?

sur une généralisation à tout le territoire. Pour mettre en place un cadre institutionnel plus adapté à la diversité de nos territoires- c'est le souhait du Gouvernement -, nous avons saisi le Conseil d'État d'un avis portant sur la différenciation des compétences des collectivités territoriales relevant d'une même catégorie et des règles relatives à l'exercice de ces compétences. Nous attendons cet avis d'ici à la fin de l'année. En fonction de cet avis, nous pourrons

TEPCV -, permettant aux territoires à énergie positive- ou TEPOS -, ces initiatives associatives et régionales, de signer une convention avec l'État et de bénéficier de financements publics. Avec le volontarisme qu'on lui connaît, la précédente ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a signé plusieurs dizaines de conventions depuis 2015, engageant l'État pour un montant prévisionnel de 750 millions d'euros. Cette dynamique est extrêmement positive pour le développement et l'aménagement durable de nos territoires et s'inscrit pleinement dans le cadre du respect des engagements pris lors de l'accord de Paris. Cependant, une circulaire du ministère de la transition écologique et solidaire du 26 septembre dernier est venue jeter un froid. ministre a admis ne disposer que de 400 millions d'euros pour les TEPCV. Plutôt que de négocier une rallonge budgétaire avec Bercy, il a donné des instructions particulièrement strictes aux préfets, le but à peine voilé étant de faire tomber un certain nombre de projets pour vice de procédure et, ainsi, défaire l'État de ses engagements. Dans mon département, l'Isère, nous estimons que la moitié des projets pourraient ainsi perdre leurs financements. Ces mesures contraignent, au-delà du raisonnable, même les projets les plus aboutis. C'est d'autant plus regrettable que la plupart des irrégularités aujourd'hui sanctionnées sont dues aux délais imposés par l'État. Non, les collectivités ne peuvent pas délibérer en quelques jours, entre l'accord de l'État sur leur programme d'actions et l'injonction de monter à Paris pour signer la convention ! Vous parliez d'État facilitateur, Je pose la question : l'État va-t-il une nouvelle fois accroître le ressentiment des collectivités locales à son égard, en réalisant des économies de courte vue, et ce dans un domaine aussi essentiel que la transition énergétique et l'aménagement du territoire, dont votre gouvernement a pourtant fait une priorité absolue ?

collectivités, dont la région des Hauts-de-France, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, et huit EPCI signataires de ce contrat de développement, qui les engage pour dix ans. Ce contrat partenarial d'intérêt national trouve sa légitimité dans les caractéristiques sociales et économiques de ce territoire, caractéristiques découlant directement de l'arrêt de la production des houillères en 1990. Le taux de pauvreté sur ce territoire de 1,2 million d'habitants est supérieur de 60 % à la moyenne nationale. Le taux de chômage oscille entre 15 % et 16 %. L'espérance de vie est inférieure de six ans à la moyenne de l'Île-de-France. Ces quelques chiffres parlent d'eux-mêmes ! La solidarité nationale à l'égard du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais est un impératif, une condition nécessaire pour que celui-ci puisse se projeter dans l'avenir et pour que ses habitants reprennent espoir. Ce n'est rien de moins que la question de la cohésion territoriale qui se joue là, pour 20 % de la population des Hauts-de-France. Aussi, monsieur le ministre, il est temps pour l'État de revenir vers les onze collectivités signataires du contrat et de confirmer ses engagements, de les « affermir », pour reprendre l'euphémisme administratif récemment entendu.

de la création de zones d'attractivité économique sur 90 % des communes du bassin minier ? La parole

devant les élus de la région, en indiquant très clairement que l'État respecterait les engagements pris sur le bassin minier. inclut la désignation du délégué interministériel, les 23 000 logements à réhabiliter et les projets de zones franches. J'y insiste, les engagements seront tenus,

pour les territoires ruraux, dont l'avenir est très inquiétant. Premier point, l'agriculture- notamment d'élevage -a perdu les deux tiers de ses emplois en vingt ans et se trouve en grande difficulté. Je souhaite que les états généraux de l'alimentation aboutissent à des solutions concrètes pour que les agriculteurs ne vendent

L'absence de médecins condamne les territoires à la désertification, compromet le retour des retraités et l'implantation des jeunes, condamne le tourisme, l'économie, les établissements

et enrayer la désertification.

dynamiques et pleins d'initiatives, en demande de financements et, surtout, d'ingénierie. Monsieur le ministre, la préfiguration de la future agence nationale de la cohésion des territoires est-elle arrêtée ? Quelle forme aura cette structure ? Quelle sera sa composition ? Quelles seront ses missions ? Quel maillage territorial assurera-t-elle ? Surtout, quels seront ses moyens ?

Vous affirmez votre volonté de renouer avec un État stratège, ce que souhaite également la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, de redonner son sens à la politique d'aménagement du territoire et de mettre en place une politique de rééquilibrage des territoires.

Doucement, mais sûrement, s'est insinuée l'idée que les compétences, les énergies, les forces vives de certains territoires pouvaient partir vers d'autres territoires, faute d'un aménagement suffisant en termes d'infrastructures, d'équipements ou de services publics ou privés. Nous avons vu grandir, s'affirmer le sentiment de déclassement et prospérer l'idée d'une France à plusieurs vitesses, se traduisant par autant de fractures territoriales, avec une myriade de territoires dont les habitants et les élus ont de plus en plus de mal à ne pas céder au découragement ou à la résignation, quand ce n'est pas à l'exaspération. L'aménagement du territoire relève pourtant prioritairement de la responsabilité de l'État, qui doit organiser, dans le cadre de la République décentralisée, des relations confiantes et bien articulées avec et entre les collectivités. La décentralisation doit signifier non pas désengagement progressif de l'État, mais « mieux d'État En se désengageant toujours plus de sa mission d'aménagement du territoire, en termes tout autant de vision que d'ingénierie, l'État a fini par laisser de nombreux territoires démunis. Or nous nous noyons encore beaucoup trop souvent sous un foisonnement de dispositifs et de politiques qui s'additionnent et se multiplient, finissant par créer de la division entre les territoires, là où il y a besoin de fluidité et d'efficacité. Ma question, monsieur le monsieur, est double. Quels sont les défis auxquels la politique d'aménagement du territoire du Gouvernement entend répondre ? Pensez-vous pouvoir conduire une politique publique efficace et cohérente dans ce labyrinthe d'acteurs et d'outils ?

Mais il faut être efficace et, donc, nous travaillons à simplifier les dispositifs. Je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons déjà répertorié plus de 1 100 dispositifs de contractualisation. Ce n'est pas raisonnable

Monsieur le ministre, le chamboulement territorial ininterrompu intervenu depuis 2010 laisse parfois penser que les gouvernants passaient plus de temps à organiser le déménagement de et dans nos territoires que l'aménagement

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous le savez comme moi, dans nos départements ruraux, le service public tient une place essentielle dans l'aménagement des territoires et son équilibre. Il contribue à structurer le territoire par une présence visible. Or, depuis quelques années, entre les réformes territoriales, les transferts de compétences, les regroupements de collectivités territoriales et, surtout, les baisses budgétaires, le service public disparaît peu à peu de nos communes et de nos cantons tribunaux, maternités, gendarmeries, trésoreries, centres de secours, services territoriaux, médicaux, postaux, bancaires, entre autres. On centralise des services qui étaient présents sur les territoires sans anticiper les fermetures et, surtout, sans concertation avec les élus. Ce mouvement engendre deux conséquences principales. D'abord, un éloignement du service public pour les citoyens. Ensuite, à moyen terme, un exode des employés des différentes structures. Ce déplacement de personnels vers des zones plus denses aboutit à des pertes indirectes pour nos territoires. ne partent pas tous seuls ; ce sont aussi leur famille et leur pouvoir d'achat qui migrent. Résultat : les élèves sont moins nombreux dans les écoles, les commerces perdent des clients et c'est toute une vie locale qui s'essouffle, ce qui anéantit bien souvent les efforts mis en oeuvre localement pour dynamiser les communes rurales.

Cet engrenage contribue donc à rendre certains territoires moins attractifs. Aider les entreprises et soutenir les investissements économiques devient alors plus complexe. Pour toutes ces raisons, il me semble indispensable de maintenir le service public dans tous nos territoires ; et, surtout, d'intégrer que notre pays pays n'est pas uniforme : la France est diverse ! Il convient que l'État apporte sa contribution à cette diversité, qui ne peut pas fonctionner uniquement avec des statistiques. Il est urgent d'imaginer des règles fiscales et sociales pour ceux qui animent nos territoires ruraux, comme, il y a quelques années, les zones de revitalisation rurale, qu'il convient de reconduire, voire de réactualiser. Avec des critères bien déterminés, une solution pourrait résider dans la création de zones franches rurales garantissant une défiscalisation totale ou partielle aux entreprises s'installant dans nos territoires défavorisés. monsieur le ministre,

vous n'avez pas eu le temps de poser précisément votre question ... Vous avez fait une déclaration programmatique à laquelle à laquelle je peux souscrire, mais qui découle d'une constatation : les services publics se sont beaucoup retirés des territoires ruraux. Là aussi, chacun pourrait en prendre pour son grade si l'on les quinze dernières années ... Nous connaissons bien la situation des services publics de l'État, y compris dans les préfectures des départements ruraux. Nombre d'agents

je tiens tout d'abord à remercier mes collègues Hervé Maurey et Louis-Jean de Nicolaÿ de leur travail, qui rappelle l'urgence de retrouver le chemin d'une politique volontariste, comme l'a dit M. le ministre, pour la constitution d'un État aménageur. Le législateur doit travailler pour que l'aménagement du territoire cesse d'être le parent pauvre des politiques publiques ! Il y a un chantier auquel je tiens et sur lequel le Sénat entend bien apporter des réponses : la revitalisation de nos centres-villes et centres-bourgs. Nos territoires connaissent un affaiblissement croissant en matière d'attractivité économique, caractérisé principalement par une importante désertification commerciale et une forte augmentation des locaux commerciaux et des logements vacants. Ce problème est devenu une question de société de première importance, car il est perceptible dans la quasi-totalité des villes moyennes et des bourgs de France. C'est pourquoi, sous l'égide du président Gérard Larcher, nous nous sommes saisis

Ainsi, nous avons suggéré, dans notre rapport publié en juillet dernier, d'envisager un moratoire national sur les implantations commerciales en périphérie, ou des moratoires locaux, ou encore des seuils d'alerte, puis de blocage en cas d'implantations trop nombreuses sur des aires géographiques données. Êtes-vous prêt, monsieur le ministre, à réfléchir avec le Sénat sur ces pistes ? Par ailleurs, sur le plan financier ou sur le plan de l'équilibre territorial, comment imaginez-vous des compensations financières ou fiscales au profit des centres-villes pour enrayer ce phénomène ? Seriez-vous prêt, par exemple, à mettre en place des zones franches

comme nombre d'entre vous, à l'intelligence territoriale et à la nécessité de faire évoluer le système en laissant la responsabilité aux élus et aux exécutifs locaux.

dans les zones périurbaines, dans cette France périphérique dont parle souvent le géographe Christophe Guilluy. Plusieurs rapports ont fait état de la dépendance réelle à l'automobile dans ces territoires périurbains et de ses conséquences sur l'exclusion de certains groupes : les handicapés, les personnes âgées, les jeunes et les ménages les plus défavorisés. Cette dépendance accentue les inégalités sociales ; elle freine les parcours professionnels et notre économie. En effet, certaines entreprises peinent à recruter pour cette raison. D'autre part, selon un rapport du Conseil économique, social et environnemental, un jeune sur trois en campagne n'a pas assisté à un entretien d'embauche faute de moyen de transport, et l'on estime à 7 millions le nombre de personnes en âge de travailler touchées par des problèmes de mobilité. Bien sûr, les innovations se font souvent dans les métropoles ou les agglomérations, où le marché est pertinent, avec une population dense, aux comportements souples et une gouvernance mieux adaptée. Pourtant, les alternatives à la voiture dans les territoires périurbains sont une véritable urgence : elles doivent être accessibles à tous, à tout moment et à moindre coût. Je pense notamment à l'autopartage, au covoiturage et au transport à la demande. Ce débat se double aussi de l'urgence environnementale, qui doit nous amener à conduire une réflexion globale sur la question des déplacements dans les zones périurbaines et rurales. Aujourd'hui, les infrastructures n'existent pas dans les territoires périurbains pour répondre à tous ces défis. Bien sûr, ce ne sont pas forcément de grandes infrastructures, coûteuses, dont nous avons besoin

Magnifique progrès en deux Républiques et 105 ans », concluait-il, avant d'ajouter : « Je ne doute pas que, le changement étant maintenant, nous allons réduire ce temps de trajet » Le changement n'étant plus maintenant, et néanmoins en marche, et le cas d'Aurillac résumant bien la situation de pans entiers du territoire et de nombreuses villes moyennes, comment comptez-vous redresser cette situation calamiteuse, pour ne pas dire scandaleuse ?

qui entend ouvrir les TER à la concurrence et supprimer les arrêts TGV dont bénéficient actuellement un certain nombre de villes moyennes, je crains que vous ne manquiez de soutien au sein du Gouvernement Pour faire un parallèle avec l'aérien, on ne dessert pas Brive avec un A380 » : voilà ce que vient de déclarer

le font ! La parole est à M. Pierre Médevielle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, en matière de téléphonie mobile, la définition des zones blanches semble totalement erronée et inappropriée. À titre d'exemple, en 2018, une seule commune de la Haute-Garonne sera définie comme une zone blanche au sens de l'ARCEP, c'est-à-dire une commune « dont le centre-bourg n'est couvert par aucun opérateur de réseau mobile

Si les opérateurs semblent toujours très satisfaits, et même plus encore, la réalité du terrain est bien différente, parfois insupportable. Il va sans dire que c'est un obstacle immense au développement de nos territoires en matière d'implantation d'entreprises et d'habitat en zone rurale. Monsieur le ministre, il est impératif de modifier les critères et les méthodes de mesure de la couverture pour disposer enfin d'un recensement conforme à la réalité du terrain. L'incitation et les supplications ayant échoué, il est nécessaire que l'État fasse preuve de beaucoup plus de fermeté pour imposer aux opérateurs privés la couverture en 3G ou 4G de l00 % de la population. Pour cela, il faut revoir les contrats d'exploitation des licences avec les opérateurs. Nous savons que vous êtes isolé au milieu de technocrates qui planchent sur la cohésion de territoires si lointains pour eux, mais cette révision se fondera-t-elle enfin sur des engagements opposables et sanctionnables, seuls susceptibles de concrétiser cette promesse du Gouvernement ?

: je vous confirme que le Gouvernement a demandé officiellement à l'ARCEP de définir un nouveau référentiel de couverture mobile. En effet, nous en avons tous assez d'entendre parler des zones blanches

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en préambule à ma question, je souhaite évoquer l'adoption, en 2012, d'une proposition de résolution du groupe du RDSE relative au développement par l'État d'une politique d'égalité des territoires. Monsieur le ministre, lorsque vous présidiez ce groupe et que vous siégiez parmi nous au sein de la Haute Assemblée, vous aviez alors déclaré qu'il fallait revenir à une certaine planification nationale, nationale, car « seul l'État peut avoir une vision globale et stratégique, ainsi que les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre l'égalité des territoires de manière concertée avec les collectivités locales ». Je partage tout à fait votre point de vue. C'est en partie la logique poursuivie par les contrats de ruralité- pendant des contrats de la politique de la ville -, dont la création par votre prédécesseur répondait à un besoin de coordination et de lisibilité des actions mises en oeuvre dans les territoires ruraux. L'Assemblée des communautés de France constate une hétérogénéité des contenus et de la qualité des contrats. Certaines collectivités qui s'attellent à élaborer une stratégie approfondie pour leur territoire et prennent le temps de la réflexion craignent de ne pas pouvoir bénéficier de ces fonds. Si la dotation de soutien

en autorisations d'engagement du programme 112, « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Cela constitue une source d'inquiétude pour les élus locaux. Aussi, je m'interroge sur la pérennité à long terme des moyens octroyés aux contrats de ruralité et sur l'avenir de ce dispositif.

Nous avons tenu à ce que les engagements de l'État puissent être honorés. C'est important pour la poursuite de ces contrats.

à une telle situation ? Parce que l'appareil d'État, cherchant à remettre en cause en permanence les lois de 1982, s'est engagé dans un processus de recentralisation forcené, et ce au mépris des des libertés locales et des élus du peuple. Et parce que l'État, pour reprendre le contrôle de la région-capitale, a créé une superstructure technocratique baptisée métropole- mot très à la mode la mode -, un monstre qui va, si nous le laissons faire, absorber demain la région, puis les départements, et sans doute après-demain nos communes. En effet, la métropolisation à marche forcée, imposée par la technostructure, est en train d'assécher totalement nos territoires et de tuer nos communes, qui sont, ne l'oublions pas, le coeur vivant de notre démocratie. C'est le cas presque partout en France : dans les communes, en région, les gares ferment, les boutiques sont moribondes, les services publics à l'abandon. Mais c'est aussi vrai dans la région d'Île-de-France, y compris dans le périmètre de la métropole, où l'on constate un désengagement de l'État et la suppression de ressources qui nous sont essentielles pour exercer nos missions, telles que la taxe d'habitation tout récemment, la baisse de la DGF, l'augmentation des péréquations, sans parler des charges transférées sans compensation.

Le développement économique se concentre autour des pôles métropolitains aux dépens des pôles d'équilibre plus modestes. C'est la réalité dans toute la France. Nos territoires ruraux sont, de fait, devenus le tiers-monde de la France, avec un flux migratoire vers les villes- ce n'étaient pas des sans-papiers, mais ils sont partis -, qui sera bientôt épuisé par manque d'habitants. Les derniers indigènes n'en peuvent plus des contraintes sans contrepartie. Ils attendent plus de souplesse ; ils attendent l'engagement du Président de la République leur permettant de prendre des initiatives. Il faut redonner

Pourtant, une politique ambitieuse d'aménagement des territoires est possible. Elle est indispensable pour notre pays

Quels sont les moyens financiers que vous envisagez de mobiliser pour faire avancer une politique d'aménagement du territoire ?

par exemple que les conseils départementaux reprochent à l'État de devoir prendre à leur charge un certain nombre de difficultés propres aux mineurs ou aux allocations de solidarité.

Monsieur le ministre, je reviens sur la question des territoires à énergie positive pour la croissance verte, car la réponse que vous avez apportée à mon collègue Guillaume Gontard me semble insuffisante. Vous Vous n'êtes pas sans connaître l'engouement de nos collectivités pour ce pertinent et structurant dispositif que l'on ne peut pas considérer comme étant une usine à gaz, pour reprendre votre propre expression. La très récente circulaire adressée aux préfets par M. le ministre d'État Nicolas Hulot prévoit en effet de réduire de 46 % les crédits de paiement du programme TEPCV, soit 350 millions d'euros des engagements pris, sur les 750 millions d'euros contractualisés sur trois ans. Première question : s'agissant de conventions pluriannuelles, il suffirait, dans les deux années à venir, de prévoir deux fois 175 millions d'euros. Les crédits inscrits à ce jour permettent d'honorer la première année d'exécution de ces conventions. Deuxième question : ne pouvant heureusement remettre en cause la signature de l'État, votre collègue propose quatre règles de gestion très contraignantes, voire dissuasives et décourageantes pour les collectivités. Il s'agit d'une remise en cause des règles du jeu. Je cite, par exemple, l'idée d'une règle de dégressivité et de pénalités de retard pour des projets au-delà du 31 décembre 2017, alors que les conventions courent sur trois années. Malheureusement, ce n'est pas qu'une idée, puisque c'est écrit dans la circulaire. Monsieur le ministre, comment comptez-vous revenir sur ces décisions et inscrire au budget les sommes correspondantes ? La

Effectivement, nous nous trouvons face à nombre d'engagements qui n'ont pas été financés ; c'est la réalité budgétaire.

intelligentes qu'elle procure. Je vous parle de confiance, celle qu'a évoquée le Président de la République envers les collectivités. La remise en cause des règles du jeu, cette méthode, je la trouve sournoise. Ce n'est rien moins que la parole de l'État qui est en question. La

Selon l'article 1 de la Constitution, la République française est indivisible. Et pourtant, il existe aujourd'hui plusieurs France. Les sociologues, les politologues, les géographes et surtout les électeurs le disent. Oui, la France est rongée par une fracture territoriale qui se révèle un des défis les plus compliqués et les plus urgents à relever : d'un côté, on l'a dit, une France dynamique, moderne, ouverte, connectée, celle des métropoles et des grandes villes, une France 2.0 qui n'a pas peur de la mondialisation et qui est armée pour l'affronter de l'autre, une France en souffrance, celle des ruralités et des périphéries, une France enracinée qui ne veut pas mourir et qui se sent déclassée, délaissée, notamment par l'État.

Mais plusieurs décisions très récentes du Gouvernement laissent sceptiques quant à sa réelle volonté de rétablir un minimum d'équité territoriale, sans parler des annulations de crédits aux collectivités : pourquoi donc avoir mis en pause le canal Seine-Nord, le barreau Picardie-Roissy et tant d'autres grands chantiers structurants et porteurs d'espoir pour nos territoires ? Par ailleurs, n'est-il pas incohérent, et même indécent, de se glorifier du dédoublement des classes de CP dans les réseaux d'éducation prioritaire alors qu'on a souvent des double ou triple niveaux à plus de vingt élèves en zone rurale ? On ne peut se satisfaire de voir des discriminations positives aggraver des discriminations négatives. Monsieur le ministre, avez-vous réellement un cap en matière d'aménagement du territoire ? Avez-vous tout simplement une boussole ?

pour la réplique. J'ai une certaine idée de la France, mais aussi de la République. La République, c'est non seulement l'égalité des droits, mais aussi l'égalité des chances, et donc un idéal d'équité territoriale. À ce titre, j'espère sincèrement que la devise qui orne les 36 000 frontons de nos mairies ne sera pas, au cours des années qui viennent, vide de sens.

Les élus locaux ont investi du temps, de l'énergie et de l'argent, en l'occurrence de l'argent public. Or les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, parce que les élus de bonne volonté se sont heurtés à la dure réalité : les médecins ne veulent pas venir, tout simplement Les fortes incitations financières ont créé une dérive insupportable. Certains effets sont désastreux. Ils aboutissent à une mise en concurrence des territoires, à ce qui pourrait s'apparenter à une perversion de l'engagement sincère au service des autres : du serment d'Hippocrate ? les personnes aux revenus modestes ; on va ponctionner les retraites au nom des économies à faire ; et on continuerait à verser des primes d'installation de 50 000 euros, à exonérer d'impôt pendant cinq ans des professionnels aux revenus plus que confortables, ayant leur patientèle toute faite dès lors qu'ils s'installent Nos concitoyens sont excédés. Ils demandent une solution rapide, efficace et durable. Rappelons que les études de médecine sont gratuites et que notre système repose sur la sécurité sociale.

il s'agit de santé publique. L'État doit protéger les citoyens et donc faire en sorte qu'il y ait des médecins et des spécialistes en nombre suffisant sur tout le territoire national. La

Certains espaces sont déjà totalement démunis. Nous ne sommes plus devant une situation d'inquiétude, mais face à une mise en danger de notre population. Le traitement classique du problème de la démographie médicale n'est plus à la hauteur de l'enjeu,

Ne pensez-vous pas que le moment est venu de le faire ? Nous avons tous déjà mis en place ces financements de structures, notamment de maisons pluridisciplinaires, annoncés dans le plan gouvernemental. S'ils sont indispensables, ces outils ne peuvent, à eux seuls, répondre au défi auquel nous sommes confrontés : un cabinet neuf sans praticien ne permet pas de soigner la population. Le plan du Gouvernement prévoit une possibilité accrue de cumul emploi-retraite pour les médecins libéraux. Cette solution en forme de compagnonnage entre générations peut permettre, à l'échelle d'un département, en synergie avec les médecins en exercice, de pallier l'urgence. Toutefois, pouvez-vous me confirmer que ces médecins retraités ne subiront aucun effet négatif administratif et financier ? Autoriserez-vous les conseils départementaux à créer des organisations de cette nature, avec l'Ordre des médecins, en veillant eux-mêmes à ce qu'aucune tracasserie administrative ou financière ne vienne frapper ces médecins de bonne volonté Enfin, une autre piste semble possible : mettre en place un service sanitaire, non pas de trois mois, comme nous avons pu l'entendre, mais d'une année, afin que les jeunes médecins puissent apporter leurs forces vives à une population aujourd'hui en abandon de soins. La parole

Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. le Premier ministre a déclaré que chaque citoyen devait avoir accès à une médecine de qualité, quel que soit l'endroit où il vit. À cet égard, l'enjeu de santé publique rejoint clairement celui de l'aménagement de notre territoire. En géographie de la santé, la question de l'inégalité dans l'accès à l'offre de soins est au coeur des débats. Mme la ministre des solidarités et de la santé a tracé les grandes lignes de sa politique qui sont de bon augure : campagnes de vaccination, lutte contre les déserts médicaux, usage de la télémédecine, S'il est un autre sujet sensible, c'est ce que l'on appelle les grandes urgences vitales, notamment cardiovasculaires. Ces dernières exigent une prise en charge rapide. À ce titre, les experts ont énoncé des recommandations sur la base des délais au-delà desquels se réduisent les chances de survie. Or, en la matière, l'inégalité territoriale existe bel et bien dans notre pays. Pour y remédier, il faut soutenir les unités de soins intensifs, investir dans des plateaux techniques appropriés et permettre aux équipes médicales spécialisées d'offrir des soins de qualité à toutes les populations. Le projet de plateau technique d'angioplastie du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui concerne 350 000 habitants, en est un exemple concret. de la santé veut, avec raison, « faire confiance aux acteurs des territoires pour construire des projets et innover dans le cadre d'une responsabilité territoriale. Cette responsabilité passe par le respect des recommandations médicales, la vie des hommes restant la première des priorités. Aussi, monsieur le ministre, je souhaite connaître les moyens que vous

La séance est levée.